nous sommes aujourd’hui réunis pour l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2025. Comme vous le savez, nous nous inscrivons dans un contexte particulier. Malgré de nombreuses heures de débats, texte en première lecture à l’Assemblée nationale s’est arrêté sans que nous soyons parvenus à son terme. Je regrette, bien sûr, que nous n’ayons pas terminé les discussions sur ces sujets fondamentaux pour les Français.

Comme nous le disons depuis le début de cette période budgétaire, et comme chacun ici le mesure, la situation de nos finances publiques exige de la responsabilité, ainsi qu’une recherche exigeante d’équilibre. La situation de nos comptes sociaux est inédite. En 2024, le déficit de la sécurité sociale dépassera de près de 8 milliards d’euros le niveau voté dans la loi de finances de la sécurité sociale initiale.

Chacun en conviendra, ce n’est pas soutenable. La situation implique des actions collectives pour y remédier. Il est de notre devoir de freiner la dépense publique ; toutes les administrations publiques doivent prendre part à cet effort. À cet égard, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 constitue une étape essentielle dans le retour progressif à l’équilibre de nos comptes sociaux. La pérennité et la préservation de notre modèle social hérité du Conseil national de la Résistance (CNR) étant en jeu, nous devons collectivement trouver une ligne de crête pour réaliser des économies sans perdre de vue les attentes considérables de nos concitoyens et leurs besoins la santé et l’accès aux soins constituent la première préoccupation des Français. C’est pourquoi ce PLFSS vise à contenir le déficit de la sécurité sociale à 16 milliards d’euros tout en finançant des mesures nouvelles. Il permet ainsi d’améliorer la trajectoire de nos comptes sociaux tout en ouvrant de nouveaux droits, au service de nos concitoyens. Je le répète, la santé des Français demeure plus que jamais une priorité de notre gouvernement ; ce budget le prouve. Nous sommes au rendez vous de ces attentes. Il s’agit d’un budget d’action pour l’accès aux soins et pour l’hôpital, qui a tant besoin de soutien. Il s’agit d’un budget de progrès, mais également de responsabilité, comme je vais m’employer à en faire la démonstration devant vous. La trajectoire d’augmentation des dépenses d’assurance maladie, c’est tout d’abord un budget de progrès. Ce budget permet de répondre à nos priorités de santé publique, comme la prévention, les soins palliatifs, la santé mentale ou l’accès aux médicaments, entre autres. L’objectif national de dépenses d’assurance maladie (Ondam) progressera, pour atteindre un peu plus de 264 milliards d’euros. C’est une hausse de 63 milliards d’euros par rapport à 2019 et de 9 milliards d’euros par rapport à 2024. Cette progression traduit concrètement notre volonté de poursuivre les investissements entrepris et de financer de nouvelles mesures attendues par les professionnels et par les patients. Cette trajectoire d’augmentation des dépenses d’assurance maladie nous permet de poursuivre la dynamique de renforcement de l’accès aux soins dans tous les territoires et pour tous. Elle permet de financer nos grandes priorités : améliorer l’organisation du système de santé, assurer le financement du système de santé, renforcer nos politiques en matière de psychiatrie et de santé mentale, travailler à l’attractivité des métiers du soin et accompagner les innovations. Nous respecterons les engagements conventionnels vis à vis des médecins, avec la revalorisation de la consultation à 30 euros dès décembre 2024. Nous poursuivrons aussi la stratégie d’« aller vers », à destination des publics précaires et éloignés du soin, en ciblant les populations des territoires sous denses. Nous développerons dans ce cadre des initiatives, comme les médicobus ou la télémédecine. Pour renforcer l’attractivité des métiers et l’accès aux soins partout, nous travaillerons, avec le concours indispensable des élus locaux, au développement des maisons de santé pluriprofessionnelles,

Les maisons de santé pluriprofessionnelles permettent aux médecins de ne plus être isolés et de créer de nouvelles synergies entre professionnels de santé. C’est un facteur d’attractivité. Ce PLFSS traduit aussi une action résolue, à laquelle je suis particulièrement attachée, en faveur des soins palliatifs : 100 millions d’euros seront dédiés à la mise en œuvre, dès 2025, de la stratégie décennale des soins d’accompagnement. Cette stratégie doit permettre dans chaque territoire le renforcement de l’offre de soins palliatifs au sein des établissements de santé et médico sociaux, mais également à domicile. La prise en charge des troubles de la santé mentale, que le Premier ministre a choisi d’ériger en grande cause nationale pour 2025, connaîtra aussi des progrès considérables. Le dispositif Mon soutien psy sera notamment renforcé, afin que chaque citoyen ait un accès simplifié et plus rapide à un psychologue, qui bénéficiera lui même d’une meilleure rémunération, et le nombre de séances prises en charge lors d’une année civile augmentera, passant de huit Les équipes mobiles psychiatrie précarité (EMPP) seront ainsi renforcées, pour aller à la rencontre des personnes les plus éloignées des soins et, surtout, de la psychiatrie. Nous le savons, prendre soin de sa santé mentale s’apprend dès le plus jeune âge : le dispositif de prévention du suicide VigilanS sera élargi aux mineurs. En outre, nous poursuivrons et amplifierons nos politiques en faveur de la prévention, en renforçant le repérage précoce. Ces actions interviendront à toutes les échelles et avec tous les acteurs, afin de prendre en charge au bon moment. Nous devons installer une véritable culture de la prévention dans notre pays ; ce budget y contribuera. Le dispositif Mon bilan prévention continuera d’être généralisé. Nous souhaitons que les mesures de prévention s’ancrent dans le quotidien de chaque Français. La part des dépenses des agences régionales de santé ciblées sur la prévention au sein de l’enveloppe du fonds d’intervention régionale augmentera de 10 %. Il s’agit d’une politique globale de la prévention que nous souhaitons faire intervenir dès le plus jeune âge,

passés devant les écrans, afin de sensibiliser les familles et de trouver des équilibres dans ces utilisations. Nous consacrerons enfin 75 millions d’euros en 2025 pour poursuivre la vaccination contre le papillomavirus au collège.

Le gain ainsi permis – de l’ordre de 256 millions d’euros – restera dans l’Ondam, au bénéfice du secteur hospitalier. Nous conforterons les mesures en faveur des soins critiques de la réforme de 2022 pour les hôpitaux, mais nous faciliterons également la gestion des ressources humaines dans les établissements de santé en travaillant particulièrement sur la régulation de l’intérim. Enfin, ce PLFSS permettra de garantir l’accès aux médicaments et produits de santé à tous les Français. La disponibilité des médicaments dans les pharmacies est un sujet de préoccupation majeur pour nos concitoyens, sur le quotidien Ce PLFSS viendra renforcer ce qui est déjà mis en place en ouvrant, par exemple, la distribution à l’unité en cas de risque anticipé de pénurie. Il prévoira aussi la possibilité de recourir à un financement dérogatoire pour des dispositifs médicaux utilisés en substitution d’un dispositif médical

Cela doit se traduire par une accentuation de la pertinence et de l’efficience de nos dépenses, de même qu’il faut amener l’ensemble des acteurs à faire preuve de responsabilité. Ils devront tous participer à la maîtrise de la progression d’une partie de ces dépenses, dans une logique d’efforts partagés et d’équité.

ailleurs, nous devrons réaliser des économies à hauteur de 5 milliards d’euros en 2025 par rapport à la progression tendancielle des dépenses. Un quantum d’efforts et des cibles d’économies ont été identifiés pour répondre à cet impératif, en respectant un effort partagé. En ce qui concerne le transfert vers les complémentaires santé,

En premier lieu, je rappelle que l’assurance maladie obligatoire finance à ce jour 80 % des dépenses de santé. Ce chiffre n’a jamais été aussi élevé dans notre pays. Il s’explique par l’effort que nous consentons chaque année pour augmenter les dépenses de santé, mais aussi par la prise en charge chaque année de 400 000 patients de plus qui basculent

qu’il en soit, c’est l’honneur de la République que de proposer à tous une prise en charge par la solidarité collective aussi élevée. Pour autant, afin de garantir la soutenabilité des finances publiques, il est essentiel de préserver cet équilibre entre l’assurance maladie obligatoire et la prise en charge par les organismes complémentaires. Pour tenir compte des positions exprimées par l’ensemble des députés et des sénateurs, le quantum a été ramené de 1,1 milliard d’euros à 900 millions d’euros. Ainsi, j’ai pu décider que le ticket modérateur de la consultation médicale, qu’il était potentiellement envisageable d’augmenter de 10 %, n’évoluera que de 5 %. La consultation médicale demeurera donc l’acte de soins de ville le mieux remboursé par la solidarité nationale. C’est essentiel pour garantir l’accès aux soins. En complément, le ticket modérateur sur les médicaments augmentera, lui, de 5 %.

Pour compenser le dérapage constaté sur les médicaments en cette fin d’année 2024 et évalué à 1,2 milliard d’euros, nous allons poursuivre le dialogue engagé avec les industriels, afin de trouver des mécanismes de contractualisation permettant de modérer les dépenses – la hausse de la clause de sauvegarde ne sera activée qu’en cas d’échec de la démarche. C’est donc dans une logique de confiance et de coconstruction que je souhaite faire au maximum face aux nouveaux défis de maîtrise de la dépense des produits de santé. Nous devons atteindre nos objectifs d’économie, mais je souhaite avant tout laisser la place à la concertation et aux débats parlementaires, comme cela a été le cas à l’Assemblée nationale.

L’examen à l’Assemblée nationale a enrichi ce projet de loi, les amendements adoptés retenus dans le texte visant à avancer sur des sujets essentiels pour la santé, notamment en termes de prévention. Je pense à l’annualisation de l’examen bucco dentaire, à la généralisation des centres de santé, à la suppression de l’adressage dans le dispositif Mon soutien psy ou encore au développement de campagnes de vaccination contre le méningocoque, qui sont autant de belles avancées pour la santé publique.

à adopter une alimentation plus équilibrée. Je sais que ce sujet tient particulièrement à cœur à Mme la rapporteure générale, Élisabeth Doineau, et à M. le sénateur Xavier Iacovelli, qui défendent des amendements en ce sens. Je ne puis malheureusement être exhaustive, mais je tiens à remercier les députés qui ont soumis des amendements et participé au débat. Aujourd’hui s’ouvre un nouveau moment essentiel du dialogue parlementaire pour la santé des Français et l’accès aux soins. J’ai été très attentive aux débats en commission, qui ont commencé la semaine dernière. J’ai écouté vos réflexions et vos propositions. Je répondrai tout au long du débat à vos interrogations et aux évolutions que vous proposez sur le texte, dans un dialogue que j’espère nourri.

pour une loi de transformation profonde de notre système de santé et de son financement. Un travail sur le temps long est nécessaire. Il nous faudra le mener ensemble, en confiance et en responsabilité. D’ici là, vous pouvez compter sur moi, tout au long de ces débats, pour rester fidèle à la méthode que je mène et que je crois juste

Je reviendrai ensuite sur la situation de nos finances publiques et de nos comptes sociaux. Je détaillerai enfin les mesures de freinage de la dépense sociale proposées par le Gouvernement pour l’année prochaine. Tout d’abord, le Premier ministre a assumé, sans ambiguïté aucune, le fait que la copie du Gouvernement était « perfectible », pourvu que la trajectoire de redressement des comptes soit respectée. Comme vous le savez, l’examen du texte n’a pu arriver à son terme à l’Assemblée nationale, faute de temps. Néanmoins, le Gouvernement a fait le choix de ne pas en revenir au texte initial, comme la Constitution l’y autorisait, mais de transmettre au Sénat un projet de loi enrichi par certaines avancées des discussions à l’Assemblée Nous avons choisi de retenir des amendements issus de toutes les sensibilités politiques, dont les dispositions constituent autant d’améliorations possibles du texte. Je pense au cumul emploi retraite des médecins, mais également aux mesures en faveur du monde agricole, à la taxation des boissons sucrées, à la réforme de la radiothérapie, à l’accès aux soins gynécologiques pour les personnes en situation de handicap ou encore à la lutte contre la fraude aux cotisations sociales. Non seulement nous sommes ouverts à la concertation avec les partenaires sociaux et aux propositions issues de vos travées, mais nous en avons surtout

Je vous confirme que le relèvement du taux de cotisation des employeurs locaux à la CNRACL sera étalé sur quatre ans, plutôt que sur trois, conformément à la proposition soutenue en commission par Mme la rapporteure générale. Nous reconnaissons en toute transparence que la copie est perfectible, pourvu que le cadre financier fixé par le Gouvernement, lui, soit bien respecté. Je tiens à saluer l’esprit de responsabilité qui a guidé les travaux de la commission des affaires sociales du Sénat, sous la présidence de Philippe Mouiller et avec la contribution de la rapporteure générale et des rapporteurs des différentes branches. À l’issue de l’examen en commission, la copie du Sénat s’inscrit pleinement dans la logique de rééquilibrage progressif des comptes sociaux proposée par le Gouvernement. Comme vous l’avez indiqué, monsieur le président de la commission, cette instance a fait de l’objectif de contenir le déficit des comptes sociaux à 16 milliards d’euros en 2025 le « premier postulat » de ses travaux. Je vous en Je vous en remercie. J’ajoute que je souscris pleinement à vos propos lorsque vous affirmez que, dès le lendemain de l’adoption du PLFSS, il nous faudra engager le temps des réformes structurelles dont notre modèle de protection sociale a besoin. rejoins les propos de Mme la ministre Geneviève Darrieussecq : ce n’est pas un PLFSS de réformes structurelles ; pour autant, il nous faudra rapidement un agenda réformateur. Le Premier ministre a d’ailleurs ouvert la voie dès vendredi dernier lors du congrès des départements de France, en annonçant un certain nombre d’évolutions dans le champ social. Ces chantiers structurels, notamment ceux qui se trouvent à l’intersection du champ social et des compétences des collectivités locales, nous engageront pour les prochains exercices. La situation de nos finances publiques, vous la connaissez. Elle exige des réponses urgentes. À l’heure où je vous parle, la dette publique dépasse les 3 220 milliards d’euros. C’est une réalité comptable. C’est surtout une réalité très concrète.

un choc d’un point représenterait en moyenne un coût de financement supplémentaire de l’ordre de 0,4 milliard d’euros. Or, comme vous le savez, pour les marchés peu importe que l’endettement soit

ce sont 60 milliards d’euros qui doivent nous permettre de contenir le déficit public à 5 % du PIB pour 2025, en vue de le ramener sous la barre des 3 % en 2029. Il s’agit au fond de préserver et d’améliorer nos conditions de financement, c’est à dire notre capacité à consolider les droits sociaux de nos concitoyens et à ouvrir de nouveaux droits, qu’il s’agisse des retraites des agriculteurs, de la prise en charge du handicap et de la perte d’autonomie, de l’indemnisation des victimes d’accidents du travail, ou encore de la prise en charge de la petite enfance. Je parle, au fond, de la capacité de notre système social à jouer son rôle de protection et de cohésion. Notre modèle, vous le savez, est fondé sur la solidarité. Ce n’est plus vrai ! C’est une valeur forte. C’est aussi et surtout une exigence de responsabilité, qui trouve sa traduction budgétaire dans le principe d’équilibre des comptes sociaux. Or cet équilibre est aujourd’hui dégradé. En 2024, le déficit de la sécurité sociale dépassera d’environ 8 milliards d’euros le niveau qui avait été voté en loi de financement de la sécurité sociale initiale. Qui gouvernait En 2025, le déficit des comptes sociaux pourrait atteindre 28 milliards d’euros sans mesure nouvelle, du fait de l’évolution spontanée des dépenses. Il y a donc un caractère d’urgence à nous engager résolument sur la voie d’un rééquilibrage des comptes sociaux. Veiller à leur équilibre, c’est tout simplement veiller à la soutenabilité de notre modèle de protection sociale. De ce point De ce point de vue, ce PLFSS marque une étape importante, mais qui en appellera d’autres. Je le dis très clairement, il faudra nécessairement que l’effort se poursuive sur plusieurs exercices

Le Gouvernement propose une progression maîtrisée de la dépense des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du fonds de solidarité vieillesse de 2,8 %, soit 18 milliards d’euros de plus, après une augmentation de 5,3 % en 2024. Sur l’année 2024, comme vous l’avez probablement lu dans la presse hier ou aujourd’hui, un risque a été détecté par la direction de la sécurité sociale sur les dépenses de médicaments, en raison d’un niveau des remises consenties par les laboratoires qui est inférieur de 1,2 milliard d’euros à la prévision qui avait été retenue jusqu’à présent. En 2024, le jeu des stabilisateurs automatiques devrait permettre de contenir environ un tiers du dépassement qui aurait résulté de cette nouvelle prévision. Ainsi l’Ondam pour 2024 sera revu de 0,8 milliard d’euros à la hausse. Le Gouvernement en a immédiatement informé le Parlement. Nous travaillons actuellement, en lien avec la commission des affaires sociales, à des mesures qui devraient nous permettre de réagir rapidement, de ramener à 0,2 milliard d’euros le dépassement par rapport à la trajectoire de l’Ondam pour 2025 présentée en texte initial. Nous proposons tout d’abord de mobiliser différents leviers de maîtrise de la dépense des médicaments, pour un rendement estimé à 600 millions d’euros. Nous proposons ensuite de baisser le plafond des remises sur les médicaments génériques, pour environ 100 millions d’euros. Nous proposons également d’introduire le tiers payant pour les médicaments biosimilaires et hybrides, afin d’accélérer leur diffusion, à l’instar de ce que nous faisons déjà pour les génériques, ce qui permettrait d’économiser 50 millions d’euros. Nous proposons encore d’activer la clause de sauvegarde sur les dispositifs médicaux. Le montant Z sera révisé à la marge, afin de tenir compte de l’actualisation des prévisions sur la base des dernières données disponibles. Cela représente 150 millions d’euros. Nous proposons enfin d’étendre les accords de maîtrise de prix volume aux transports sanitaires. Cela représente 100 millions d’euros d’économies, soit l’équivalent du dérapage constaté en 2024 pour cette dépense. Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, en toute transparence, les mesures que propose le Gouvernement

ainsi, les amendements déposés en vue d’autoriser l’assurance maladie à appliquer de nouveaux plafonds de franchises spécifiques pour les transports sanitaires, d’une part, et les dispositifs médicaux, d’autre part, recevront un avis favorable. Compte Compte tenu des délais de mise en œuvre opérationnels de ces dispositifs, il n’en est cependant pas attendu d’économies significatives dès l’année prochaine. En 2025, quatre piliers permettront de ramener le déficit de la sécurité sociale à 16 milliards d’euros, tout en finançant des mesures nouvelles. premier pilier est la modulation de l’indexation des pensions de retraite. Comme cela a été annoncé, un compromis a été trouvé, afin de corriger la copie initiale présentée par le Gouvernement – c’était d’ailleurs l’une des propositions de la commission des affaires sociales du Sénat. Toutes les retraites feront l’objet au 1 janvier 2025 d’une revalorisation égale à environ la moitié de l’inflation. Les petites retraites feront l’objet d’une revalorisation complémentaire à l’été pour qu’elles ne soient pas affectées par cette mesure. Je précise que le calendrier et les modalités de revalorisation des minima sociaux restent inchangés. Le deuxième pilier est la maîtrise des dépenses de l’Ondam, qui permettra de ramener la progression de celui ci à son niveau spontané de 2,8 %. Les marges de manœuvre que nous dégageons nous permettront de financer les mesures nouvelles que le Gouvernement souhaite déployer : en faveur des professionnels de santé libéraux, que nous proposons de revaloriser une enveloppe de 1,6 milliard d’euros ; en faveur de l’hôpital, dont nous proposons d’augmenter le budget de 3 milliards d’euros en faveur des établissements sociaux et médico sociaux, dont nous proposons d’accroître le budget de plus de 2 milliards d’euros. Le troisième pilier est constitué par les réformes d’efficience. Je pense notamment à celle des allégements généraux, qui doit nous permettre de lutter plus efficacement contre les trappes à bas salaires. Mais, comme vous le savez – nous l’avons dit à plusieurs reprises –, nous sommes ouverts à des ajustements sur ce point, afin de modérer la contribution demandée aux entreprises et aux employeurs. pilier – que nous continuerons à amplifier nos efforts en matière de lutte contre la fraude sociale, en lien avec les caisses du régime général, l’Urssaf et la Je l’ai dit, nous avons repris plusieurs amendements en ce sens qui étaient issus de l’Assemblée nationale. Je relève également des propositions intéressantes de la commission des affaires sociales du Sénat sur ce sujet. Mesdames, messieurs les sénateurs, je me réjouis, aux côtés de mes collègues du Gouvernement, de travailler avec vous dans les prochains jours pour améliorer encore ce PLFSS, qui est avant tout, je le crois profondément, un texte d’urgence, mais aussi et surtout de responsabilité collective. La parole

le travail est au cœur du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le travail finance notre protection sociale : les contributions sur le travail sont encore la ressource

Notre discussion s’ouvre aujourd’hui dans un contexte différent, dans un environnement économique qui se tend, avec un niveau élevé de défaillances d’entreprises et d’importantes conséquences sociales dans les territoires, avec l’annonce de plusieurs plans sociaux. Je profite de ce passage à la tribune pour saluer les projets d’accords trouvés vendredi dernier entre les organisations de salariés et les organisations patronales sur l’assurance chômage et l’emploi de seniors. Ce premier succès démontre qu’une nouvelle méthode et un dialogue social renouvelé permettent des avancées importantes. Il souligne également combien les partenaires sociaux sont des acteurs incontournables de la vie démocratique, sociale et économique du pays.

Pour tous les salariés de ce pays, pour tous les employeurs, nous avons la responsabilité collective de protéger notre modèle social, de le rendre plus efficace et d’en garantir la soutenabilité. Si le travail et l’activité financent notre protection sociale, aujourd’hui, objectivement, ils ne suffisent pas. Nous devrons, à terme, réfléchir à un mode de financement différent de notre protection sociale. Dans l’immédiat, personne ne peut se satisfaire que notre modèle social soit financé par le déficit et l’emprunt Il nous faut donc travailler plus et mieux, tous et mieux, plus longtemps et en meilleure santé, afin de financer nos investissements d’avenir et notre protection sociale. Ministre du travail et de l’emploi, mon rôle est d’abord de faire en sorte que notre économie sorte que notre économie continue à créer des emplois. Il est aussi de faire en sorte que ces emplois offrent un travail de qualité, exercé dans de meilleures conditions et que cette contribution soit reconnue. C’est ce que nous proposons aussi au travers de ce PLFSS. Sur l’emploi et le travail, le PLFSS est d’abord un outil pour favoriser le dynamisme salarial et le travail qui paie. C’est le sens premier de l’article 6. Nous avons un double impératif : soutenir l’emploi dans le contexte particulier que l’on connaît ; développer la compétitivité de nos entreprises. Avec cet article 6, nous souhaitons ouvrir un débat important.

Je suis persuadée qu’il ne peut pas y avoir de cohésion sociale sans entreprises qui marchent, et inversement. La préservation de l’emploi est une priorité ! Je partage donc le souci de protéger l’emploi et de limiter la dynamique d’augmentation du coût des allégements généraux. Pour tenir compte de ces différentes contraintes, le Gouvernement, comme Laurent Saint Martin l’a récemment souligné, est prêt à revoir le rendement de cette mesure. Ce sera tout l’objet des discussions que nous aurons au Sénat. Nous devrons également avancer sur l’articulation entre salaires, cotisations sociales et prestations. C’est l’un des enjeux de l’allocation sociale unique, chantier que le Premier ministre vient de relancer, sous l’égide de mon collègue Paul Christophe. De la même manière, du PLFSS, sur les minima conventionnels et les classifications professionnelles, qui contribuent grandement au tassement des grilles salariales, nous avons commencé à recevoir les branches qui tardent trop et, de façon structurelle, à négocier sur ces points.

La proposition du Sénat tendant à instituer une contribution de solidarité par le travail est intéressante. Elle permettrait de mieux financer la branche autonomie, tout en présentant une grande souplesse d’application, laissant de la place au dialogue social. concerne les pensions de retraite, votre commission des affaires sociales a adopté une nouvelle rédaction de l’article 25, avec une revalorisation en deux temps : de l’ordre de la moitié de l’inflation pour tous au 1 janvier et une revalorisation complémentaire rétroactive à intervenir au 1 juillet, de manière que les pensions inférieures au Smic soient revalorisées au niveau de l’inflation. Je veux rappeler ici pourquoi nous soutenons cette mesure. Nous partageons tous l’objectif de garantir la soutenabilité et la pérennité de notre régime de retraite par répartition. La dégradation de la situation économique appelle des mesures qui produisent leur effet à court terme, tout en gardant un esprit de solidarité et de justice.

Enfin, garantir la soutenabilité du système de retraite oblige aussi à regarder en face la situation de certains régimes déficitaires, comme la CNRACL. Le régime des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers souffre d’une démographie défavorable, avec moins de cotisants, plus de pensionnés et un taux de cotisations employeur très inférieur à celui du reste de la fonction publique. Sans réforme, la CNRACL présenterait, en 2030, un déficit de 10 milliards d’euros – sur les 14 milliards d’euros de déficit de l’ensemble de la branche vieillesse. Nous y répondons en procédant à une augmentation progressive des cotisations des employeurs. Nous avons fait le choix de hausses graduelles, plutôt que du choc préconisé par les inspections dès 2025. Les discussions en commission des affaires sociales ont permis d’enrichir ce texte, et les dispositions de l’amendement déposé par Mme la rapporteure

J’ai conscience qu’il s’agit d’une réponse de court terme, qui transfère le coût vers l’employeur et qui risque de polariser un peu plus encore le monde du travail, entre les salariés qui sont protégés par de bonnes conventions collectives et ceux qui ne le sont pas. Cette mesure comptable était nécessaire, sans être satisfaisante. Nous devrons impérativement réexaminer le système des IJ dès que le budget sera voté, afin de trouver un meilleur équilibre, plus juste, entre responsabilité individuelle, responsabilité de l’entreprise et solidarité nationale. Je souhaite que nous puissions en discuter au Parlement, mais nous devrons aussi échanger avec les partenaires sociaux et les chercheurs en mettant ces sujets sur la table dès janvier 2025. Après le travail qui paie et la responsabilité budgétaire, un troisième grand axe de ce PLFSS pour le travail et l’emploi est formé de mesures de justice sociale et d’appui aux entreprises. En matière agricole, ce PLFSS contient plusieurs progrès significatifs, comme la pérennisation de la hausse des exonérations de cotisations patronales sur le travail saisonnier et la hausse des exonérations de cotisations au moment de l’installation, des avancées qui ont été demandées en janvier dernier. concerne les exonérations pour les travailleurs saisonniers, nous avons complété le dispositif : à l’Assemblée nationale, nous avons pu avancer avec les députés engagés sur ce sujet, de manière à neutraliser les effets de la réforme des allégements généraux sur le dispositif

a déjà été présenté aux sénateurs et députés ultramarins. Ce bilan montre qu’il existe des marges d’efficacité pour que cette exonération soit mieux ciblée et plus efficace et pour qu’elle soutienne mieux l’emploi. Un travail doit être engagé sur le sujet dans le cadre de l’ordonnance prévue à l’article 6.

disposition permet la bonne transposition dans la loi de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 15 mai 2023 concernant l’indemnisation des accidents du travail. Je sais que le Sénat y est particulièrement attentif – je pense notamment aux sénatrices Annie Le Houerou et Marie Pierre Richer, qui ont rendu un rapport d’information sur la question au début du mois d’octobre. La transposition est un exercice délicat : le passage

Cet automne, un travail soutenu, réalisé avec les partenaires sociaux et les parlementaires, a permis d’aboutir à une meilleure transcription de l’ANI, une transcription plus complète qui apporte des améliorations substantielles.

douloureuses, celles de personnes qui n’ont plus qu’une faible espérance de vie et qui préfèrent opter pour une sortie en capital, avec de l’argent immédiatement disponible, plutôt que pour une rente. C’est ce qui sera rendu possible par l’article

Beaucoup de discussions ont lieu depuis que le texte est passé en conseil des ministres. Certains débats ont commencé à l’Assemblée nationale sans pouvoir aboutir. Il vous revient maintenant de faire des choix pour soutenir le travail et l’activité, des choix responsables et qui ne cèdent en rien au court termisme. La parole

nous avons ensemble une responsabilité sur la partie du PLFSS qui concerne les solidarités. Comme vous le savez, l’Assemblée nationale n’a pu aller jusqu’au bout de l’examen du texte proposé.

Je rappelle également que le texte qui vous est proposé a été préparé dans un cadre budgétaire contraint, et rapidement. Il est donc perfectible. Je sais que vous avez des avancées importantes à proposer ; j’y reviendrai. nous avons eu le temps de les évoquer en audition, je tiens à rappeler ici les grands principes qui guident le budget de mon ministère, à savoir l’efficience, qui va de pair avec la fraternité, avec un budget d’investissement dans notre avenir, c’est à dire dans notre modèle de solidarité, et la prise en compte de notre transition démographique. Dans le contexte budgétaire actuel, nous savons que les plus vulnérables d’entre nous seraient les premiers à souffrir d’un dérapage des finances publiques. Les commissaires des affaires sociales peuvent en témoigner compte tenu des échanges mon ministère entend prendre toute sa part à l’effort collectif pour que la fraternité – la troisième valeur républicaine, celle qui apporte une indispensable dimension humaine – continue d’être un principe général d’action publique. Je les remercie du travail qui a été mené. Celui ci sera encore approfondi à partir d’aujourd’hui dans cet hémicycle. En effet, si les moyens des solidarités sont en hausse pour accompagner toutes les familles et tous les Français, il nous faut aussi – c’est indispensable – renforcer l’efficacité au juste coût, autrement dit l’efficience de nos moyens publics. nous encouragerons les améliorations dans les pratiques d’achat des établissements et les mises en commun des ressources. Nous favoriserons une sobriété médicamenteuse dans les établissements, car nous savons qu’un usage abusif des médicaments peut détériorer la santé et altérer la qualité de vie de nos concitoyens.

Je commencerai en évoquant la politique familiale, qui est une priorité du Gouvernement et du Premier ministre. Ce PLFSS conforte tout d’abord les moyens prévus pour le service public de la petite enfance. Celui ci est crucial et a un impact considérable sur la vie des Français. Il est nécessaire d’agir de manière résolue et continue si l’on veut réduire les tensions sur l’offre d’accueil et la charge qui en découle pour les parents, et nous devons aller plus loin dans le contrôle de la qualité de cette offre. Concrètement, nous renouvelons le défi de créer 35 000 places dans les établissements d’accueil du jeune enfant, en finançant les investissements nécessaires à horizon de 2027. Nous poursuivons également la revalorisation des professionnels, qui sont essentiels à notre ambition pour la petite enfance. Dès cette année, le bonus attractivité commence son déploiement, pour augmenter les salaires nets à hauteur de 150 euros en moyenne en début de carrière. Le service public de la petite enfance bénéficiera à partir du 1 janvier 2025 d’un nouvel élan, grâce aux compétences obligatoires conférées aux communes : celles ci auront le rôle de recenser l’offre disponible et disposeront enfin de nouveaux outils pour assurer la qualité de l’accueil du jeune enfant. fait, l’objectif de ce service public est aussi et surtout de renforcer la sécurité des jeunes enfants. Les lieux d’accueil sont les premiers lieux de la vie ; ils doivent la protéger. Nous devons tourner la page des intolérables situations d’optimisation financière, qui font souffrir nos enfants et les professionnels et qui créent une défiance des parents. Rôle renforcé des communes, revalorisation des professionnels, création de nouvelles places : telles seront les clés d’une confiance retrouvée et d’un secteur consolidé.

que nous devons toutes et tous ici prêter une attention particulière aux familles monoparentales, dont la charge incombe plus souvent à des femmes. À partir de 2025, comme prévu, la branche famille financera à hauteur de 600 millions d’euros en année pleine une réforme du complément de libre choix du mode de garde.

Nous allons reprendre les concertations pour faire plus simple et plus efficace, au service du développement lors des 1 000 premiers jours de l’enfant et de l’égalité entre les femmes et les hommes. La valeur de fraternité porte également nos actions en faveur des personnes en situation de handicap. Je souhaite, avec Charlotte Parmentier Lecocq, conforter les mesures de la Conférence nationale du handicap (CNH) et la dynamique impulsée par les jeux Paralympiques en faveur d’une société plus inclusive. Le PLFSS prévoit ainsi une accélération du déploiement des 50 000 nouvelles solutions d’accompagnement. Le rythme prévu s’appuyait sur 200 millions d’euros environ par an. Nous porterons l’enveloppe disponible à 270 millions d’euros supplémentaires en 2025. Cette dynamique doit rendre possible, dès 2025, le déploiement effectif de 15 000 solutions plus individualisées, plus adaptées aux besoins spécifiques des personnes, au plus près de leurs lieux de vie. On ne peut pas tout standardiser. Nos politiques visent à faciliter le sur mesure. Si besoin, ces solutions pourront bénéficier, en complément, du fonds de transformation de l’offre de 250 millions d’euros annoncé en Comité interministériel du handicap et confirmé dans le PLFSS. La transformation vers le milieu ordinaire ne se décrète pas. Elle s’accompagne et doit être dotée de moyens. Dans ce contexte, nous aurons une attention particulière à l’école pour tous, à laquelle je crois profondément.

Une société est véritablement inclusive quand elle combat activement les préjugés dès le début de la sociabilisation. C’est de cette manière que l’on bâtit une société nativement inclusive. Pour ce faire, notre école a besoin de moyens d’accompagnement médico sociaux. Mon ministère est en mesure de les fournir.

c’est à dire 6 ans et 344 jours, et non 5 ans et 344 jours. Cette correction a son importance, car un repérage et un diagnostic précoces sont essentiels pour éviter les risques de surhandicap. J’en viens à un sujet d’attention pour lequel les défis sont toujours devant nous : le vieillissement de la population. Nous en avons beaucoup parlé, et nos préoccupations sont communes. Oui, il faut se préparer dès maintenant à l’augmentation importante du nombre de personnes de plus de 85 ans qui auront besoin d’un soutien dans leur autonomie.

En anticipant ce phénomène et en repensant notre approche politique, nous ne ferons pas seulement face à cette situation : nous garantirons également la préservation des valeurs fondamentales qui font la France. Dans l’immédiat, nous faisons face à une urgence : la situation financière difficile des Ehpad ne peut plus durer C’est dans l’intérêt des résidents, des professionnels, des familles et des valeurs sociales de notre pays. Aujourd’hui, 90 % des Ehpad de demain sont déjà là. Nous avons besoin d’eux ! Or leurs difficultés financières sont structurelles, comme l’ont montré plusieurs rapports parlementaires.

Certains logent des étudiants, abritent des crèches conjointes, des services publics. Certains accueillent même parfois des lieux de convivialité pour tout un quartier. Des investissements immobiliers supplémentaires sont prévus à cet effet dans le PLFSS. Évidemment, le financement des Ehpad doit également être simplifié. Ils ne sont pas uniquement financés, comme vous le savez, par la sécurité sociale. Or le renvoi de responsabilités entre cofinanceurs est délétère. En complément d’une mesure de la loi Bien Vieillir, le PLFSS prévoit ainsi de financer de manière volontariste l’expérimentation du financement de l’entretien de l’autonomie en Ehpad, qui relève aujourd’hui des départements, par la branche de la sécurité sociale du même nom. Cette réforme, pour laquelle 23 départements candidats sont retenus, représente un surcoût total d’environ 200 millions d’euros pour la sécurité sociale. nous croyons tous au caractère structurant de cette expérimentation, au point que certains voudraient en réduire la durée de quatre à deux ans. C’était le souhait de la députée Annie Vidal, que je me permets de citer ici. Je comprends que c’est aussi votre souhait, madame la sénatrice Deseyne.

augmenteront, tous départements confondus, le recrutement d’environ 6 500 professionnels supplémentaires, pour atteindre au plus vite les 50 000 équivalents temps plein (ETP) supplémentaires annoncés pour 2030. Ces évolutions aboutissent à une hausse des moyens dédiés aux personnes âgées d’environ 6 % en soit une augmentation supérieure à celle de l’année dernière. Accompagner le vieillissement, c’est également soutenir nos aides à domicile, grâce auxquelles se réalise le souhait de nombreux Français de vieillir chez eux, que ce soit à leur domicile historique ou dans une résidence adaptée. En accord avec la loi Bien Vieillir d’avril 2024, nous proposons, dans ce PLFSS, une nouvelle aide financière de 100 millions d’euros à destination des départements, qui la dirigeront vers les aides à domicile, afin de soutenir une partie de leurs dépenses en mobilité. qui sont souvent des femmes, financent encore leurs déplacements professionnels, ce qui est inacceptable ! Surtout, et c’est un effort important annoncé par le Premier ministre lors des Assises des Départements de France en fin de semaine dernière, nous allons préserver intégralement les taux de compensation des départements sur les dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie et de prestation de compensation du handicap en 2025. Cela a un coût : environ 200 millions d’euros. Cette somme sera ajoutée aux dépenses de la branche. Mais c’est aussi un signal fort

C’est ce que nous faisons avec ces 200 millions d’euros pour 2025, en nous assurant que, malgré une hausse dynamique des dépenses liée au vieillissement, le taux de compensation sera maintenu. En lien avec Départements de France et à partir de ce premier mouvement significatif, nous négocierons ensemble des règles d’évolutions claires en 2026 et pour les années suivantes, afin de faire converger les taux de compensation et de donner à ces collectivités essentielles une visibilité sur l’accompagnement à venir de la sécurité sociale par rapport à des besoins en hausse. C’est aussi cela la nouvelle méthode partenariale du Gouvernement avec les collectivités territoriales sur cet enjeu déterminant du vieillissement. je souhaite conclure en évoquant un sujet que je porte depuis plusieurs années, celui des 11 millions d’aidants de personnes en situation de handicap ou âgées en perte d’autonomie. Je vous confirme que le PLFSS prévoit une augmentation des moyens pour le déploiement de nouvelles places de répit, et je surveille avec attention le déploiement des droits rechargeables du congé proche aidant pour chaque nouvelle personne aidée. Je souhaite par ailleurs donner un nouveau souffle à la stratégie Agir pour les aidants, que les récents soubresauts démocratiques n’ont pas permis de porter autant que ce sujet le méritait. Un comité de suivi aura bien lieu avant la fin de l’année. J’en profite pour ajouter que, dans une logique de convergence sociale à Mayotte, madame la sénatrice Ramia, et d’égalité de traitement entre tous nos concitoyens, je serai favorable à l’extension de l’assurance vieillesse des aidants à Mayotte.

de l’aventurisme juridique, donc financier, dès lors qu’une sécurité sociale en fort déficit se finance en empruntant à court terme sur les marchés. J’en viens aux mesures de redressement proposées par le Gouvernement dans la sphère sociale. Les chiffres sont sans précédent : 14,8 milliards d’euros pour l’ensemble des administrations publiques et 12,4 milliards d’euros pour la seule sécurité sociale. La nécessité de mesures d’une telle ampleur apparaît dans le seul fait que, malgré leur montant, elles ne suffiraient pas à ramener le déficit sur la trajectoire prévue il y a un an.

d’abord, il ne faut pas dégrader un solde déjà très préoccupant, ce qui suppose, même si c’est difficile et, je le dis à titre personnel, douloureux, des efforts de tous.

afin d’étaler davantage l’effort des collectivités locales et des hôpitaux. Nous comptons aussi sur un geste du Gouvernement en faveur des Ehpad et des départements pour l’aide à domicile. La sagesse enjoindrait également de ne pas baisser de dix points le ticket modérateur sur les consultations médicales.

Elle dégagerait aussi des fonds pour des mesures nouvelles, comme la réforme de la prise en charge des fauteuils, qui a été annoncée par le Président de la République en début d’année, mais qui n’avait toujours pas trouvé son financement…

Pour moi, comme pour chacun d’entre vous, ce qui compte avant tout, c’est de maintenir notre protection sociale au plus haut niveau. Mais nous n’y parviendrons pas si nos finances publiques cessent d’être soutenables. Nous devrons donc être prudents et courageux. Ce sera Ce sera certainement douloureux, mais le pire serait de n’avoir ni la volonté ni le courage de formuler des propositions à la hauteur des enjeux. La

Alors que le déficit se creusera encore au moins jusqu’à 2028, l’horizon d’un retour à l’équilibre s’éloigne durablement, nous rendant particulièrement vulnérables à tout nouveau choc conjoncturel.

Le Gouvernement nous informe que la situation en 2024 serait plus dégradée encore que ce qui était anticipé. Au pied du mur, nous n’avons d’autre choix que de tenir compte de ces nouveaux éléments de contexte pour 2025. l’Ondam atteindrait 264 milliards d’euros, en hausse de 2,6 % par rapport à l’exécution de 2024. Cette projection, fortement contrainte, imposerait un niveau d’économies sans précédent, notamment sur les soins de ville et les produits de santé.

En deuxième lieu, il convient de limiter autant que possible la hausse du ticket modérateur annoncée par le Gouvernement sur les consultations de médecins et de sages femmes. Celle ci constitue un report de charges vers les assurés et induit une privatisation du financement de ces actes pivots.

La situation, alarmante, exige une mobilisation collective pour dessiner les contours d’un redressement financier dans un horizon raisonnable, sans sacrifier aux nécessités du présent. C’est à la recherche de cet équilibre délicat que nous invite le PLFSS : tenir des objectifs de dépenses resserrés tout en continuant à œuvrer pour la santé des Français. Parce que ce texte impose à tous les contribuables des efforts considérables, l’inaction face à la fraude sociale et à l’inefficience de la dépense serait inaudible, voire coupable. La commission a donc adopté deux amendements visant à renforcer notre arsenal de lutte contre la fraude, en sécurisant la carte Vitale et en organisant une meilleure articulation avec les complémentaires santé. Elle a également cherché à améliorer la pertinence des dépenses de santé, en limitant les actes redondants par la consultation et l’alimentation du dossier médical partagé

Ce type de mesures doit demeurer exceptionnel et nécessiter une autorisation parlementaire. Nous vous inviterons également à recentrer la procédure d’accompagnement à la pertinence des prescriptions sur les produits de santé et les actes pour lesquels elle est la plus utile. Dans le contexte actuel, il serait particulièrement inacceptable de réduire le temps médical disponible par l’ajout de formalités inutiles. La commission formulera, par ailleurs, plusieurs propositions destinées à améliorer l’anticipation et la gestion des pénuries de médicaments,

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, une stratégie de financement à la fois crédible et soutenable est désormais impérative. Cet effort exige des arbitrages difficiles, dès 2025, ainsi que des choix politiques assumés. La commission invitera le Sénat à y prendre sa part, tout en demeurant attentif aux besoins de santé des Français. La parole

Au delà de ces dépenses ponctuelles, le solde de la branche vieillesse resterait fortement déficitaire pour les années à venir, en raison de l’augmentation du nombre des retraités et de la diminution de la population active. Les effets de la réforme des retraites seront au rendez vous, puisque celle ci rapporterait 8 milliards d’euros en 2028. Ils ne seront toutefois pas suffisants pour ramener la branche vieillesse à l’équilibre. Aussi, je crains que nous ne soyons contraints, à l’avenir, de porter d’autres réformes des retraites.

Il nous faut désormais assainir nos finances, afin de ne pas porter préjudice aux générations futures et de préserver nos acquis sociaux. Je souhaite toutefois que ces efforts soient répartis avec équité

que je défendrai. En outre, la commission propose que, exceptionnellement, les pensions de retraite ne soient pas revalorisées au 1 janvier au niveau de l’inflation de l’année passée, mais à hauteur de la moitié de la hausse Nous demandons à nos concitoyens retraités de consentir à cet effort après la forte revalorisation dont ils ont bénéficié l’an dernier. Nous ne sommes néanmoins pas égaux face à l’inflation ; il faut pouvoir se nourrir et se loger décemment.

puisse être rachetée par la Cades. Enfin, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale comprend la réforme très attendue du calcul de la retraite de base des non salariés agricoles sur les vingt cinq meilleures années d’assurance.

elle exclura du calcul les mauvaises années de récolte et augmentera les pensions des polypensionnés, qui sont 85 % des non salariés agricoles. Les monopensionnés aux revenus les plus faibles ne seront pas perdants, grâce au rattrapage des de pension, dont les non salariés exerçant leur activité agricole à titre secondaire pourront désormais bénéficier.

Je souhaite que cela soit acté. Mes chers collègues, ces mesures donneront lieu à des débats riches et fournis. J’ai à cœur, néanmoins, que nous concilions nos deux objectifs de réduction de nos dépenses et de protection du pouvoir d’achat des citoyens les plus fragiles.

ait été mise en place sur la période. Selon les prévisions, la branche serait même en déficit de 500 millions d’euros en 2026. La période de la covid de 2020 exceptée, ce serait une première depuis 2018. Bien que les prévisions pluriannuelles laissent entrevoir un retour ultérieur à un excédent budgétaire, la commission s’interroge sur la capacité de la branche à répondre aux nombreux défis auxquels elle devra faire face dans les prochaines années.

au contraire, une chance pour entamer ou reprendre des travaux sur les réformes structurelles nécessaires à la relance de la natalité dans notre pays : création d’un véritable congé de naissance, réforme du financement des établissements d’accueil du jeune enfant – comme l’a dit M. le ministre des solidarités –, ou encore véritable universalité des allocations familiales.

trajectoire inquiétante : alors que le désir d’enfant des Françaises et des Français serait de 2,4, l’indice conjoncturel de fécondité s’est établi, en 2023, à 1,68, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale.

Oui, mes chers collègues, il y a urgence à promouvoir une politique familiale ambitieuse et refondée ! La parole

Cette situation résulte d’une faible dynamique des recettes, accentuée par les de taux avec la branche vieillesse en 2024 et en 2026, et conjuguée à des dépenses qui continuent de progresser, alimentées par l’accroissement du poids des transferts – j’y reviendrai –, mais également par des améliorations notables de la réparation et par une politique de prévention plus ambitieuse. Il convient de saluer l’ébauche du virage préventif tant attendu par les partenaires sociaux et la commission, stimulé par la montée en charge des mesures adoptées lors de la dernière réforme des retraites et par la hausse des moyens attribués, dans la nouvelle convention d’objectifs et de gestion (COG), au Fonds national de prévention des accidents du travail

Après le fiasco de l’article 39, les partenaires sociaux ont su maintenir le dialogue pour aboutir, par la négociation, à une réforme pragmatique et équilibrée, pour une politique de réparation plus juste. Conformément à leur volonté, la rente viagère et l’indemnité en capital présenteront, désormais, une nature duale retranscrite dans leur mode de calcul. Une part fonctionnelle s’ajoutera donc au montant actuel des prestations, qui deviendra leur part professionnelle. Il en résultera, pour tous les futurs bénéficiaires, une revalorisation représentant, à terme, un effort bienvenu de 500 millions d’euros pour la branche. La commission, fidèle à la position exprimée par la mission d’information, a soutenu ces dispositions tout en veillant à ménager un équilibre spécifique pour les victimes de faute inexcusable de l’employeur, en renforçant leur indemnisation indemnisation de court terme. Afin que leurs préoccupations propres soient entendues, elle a également souhaité impliquer davantage les associations de victimes à la conception des textes d’application nécessaires au déploiement de la réforme, tout en respectant le cadre paritaire et le rôle primordial des partenaires sociaux dans le processus. Comme elle l’avait fait l’an dernier, la commission appelle enfin le Gouvernement à retranscrire sans délai le reste du contenu de l’ANI. Plus de dix huit mois après la signature de cet accord, les mesures ambitieuses préconisées par les partenaires sociaux en matière d’aide humaine et de prévention ne sauraient être mises de côté plus longtemps. Vous l’avez compris, mes chers collègues : la trajectoire de la branche AT MP marque, pour les années futures, un effort considérable pour la réparation et la prévention. C’est pourquoi je vous inviterai à adopter l’article 28 fixant l’objectif de dépenses de la branche à 17 milliards d’euros pour 2025, afin de dégager un excédent de 200 millions d’euros. J’en viens à la question épineuse des transferts, principaux responsables de la dégradation de la situation financière de la branche. En effet, un euro sur six perçus par la branche AT MP est reversé à d’autres entités. Le transfert à la branche maladie atteindra 2 milliards d’euros à l’horizon 2027, afin de prendre en compte la révision à la hausse de l’estimation du coût de la sous déclaration par la commission. Dès 2025, le transfert augmentera de 400 millions d’euros, pour un montant total de 1,6 milliard d’euros. J’ai auditionné le président de cette commission. Il m’a donné des garanties sur la sincérité de son mode de calcul, qui prend également en compte la surdéclaration des AT MP. En outre, force est de constater que la branche s’apprête à fournir un effort inédit depuis le retour aux excédents en faveur de la prévention et de la réparation.

ne défendra pas d’amendement visant à diminuer le niveau du transfert au titre de la sous déclaration. Estimant que la branche AT MP n’a pas à servir de variable d’ajustement pour combler le déficit des autres branches, la commission s’opposera toutefois sans ambiguïté, dans les années futures, à toute augmentation des cotisations AT MP induite par la hausse du transfert au titre de la sous déclaration. Enfin, la dotation de la branche AT MP au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) représentera près d’un demi milliard d’euros en 2025 – elle aura doublé en deux ans. Dans ce contexte, je regrette que l’État n’ait pas augmenté sa subvention d’un centime, bien que celle ci ne couvre pas, tant s’en faut, les dépenses qu’il est censé prendre en charge au titre de la solidarité nationale. J’appelle donc de nouveau solennellement le Gouvernement à rééquilibrer l’effort financier en faveur du Fiva, pour que l’État prenne enfin sa juste part. Je me réserve le droit de déposer, l’an prochain, des amendements en ce sens si la situation n’évolue pas. La parole est à Mme le rapporteur.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, malgré le contexte budgétaire que nous connaissons, ce PLFSS s’évertue à préserver la branche autonomie. L’objectif de dépenses pour 2025 s’élève à 42,4 milliards d’euros. Il est en augmentation de 6 % par rapport à l’année 2024 et intègre une hausse de 4,7 %, à champ constant, à l’Ondam relatif aux établissements et services médico sociaux. Le dynamisme des dépenses permettra principalement de financer la montée en charge de mesures récentes. Celles ci n’ont pas de traduction dans le PLFSS, puisque leur mise en œuvre relève du domaine réglementaire. Dans le champ du grand âge, 6 500 recrutements sont prévus dans les Ehpad. En outre, un fonds de 140 millions d’euros sera déployé pour accompagner la transformation des établissements et soutenir les Ehpad ultramarins. La reconduction du fonds d’urgence de 100 millions d’euros pour les établissements et services en difficulté n’est pas envisagée. Il est vrai qu’un fonds d’urgence n’a pas vocation à perdurer et que l’effort doit porter sur des mesures structurelles. Pour autant, nous devons rester vigilants à l’égard des structures qui sont au bord de la fermeture. Dans le champ du handicap, peu d’annonces ont été faites. En 2025, 15 000 nouvelles réponses médico sociales devraient être développées pour les personnes en situation de handicap, dans le cadre du plan de création de 50 000 solutions à horizon 2030.

Finalement, dans ce PLFSS, seul un article relève de la cinquième branche. Il concerne l’expérimentation sur le financement des Ehpad et des unités de soins de longue durée que nous avons votée l’année dernière. À partir du 1 janvier 2025, dans les départements volontaires, les sections de financement soins et dépendance seront fusionnées sous l’égide des ARS. À l’article 21, le Gouvernement propose d’augmenter de 20 à 23 le nombre des départements qui pourront prendre part à l’expérimentation. Il précise aussi les dispositions financières relatives au dispositif. Face à l’engouement des départements, l’augmentation du nombre de participants est évidemment une bonne nouvelle. De fait, la simplification du régime de financement des Ehpad est très attendue par le secteur. Je vous proposerai donc de réduire la durée de l’expérimentation de quatre ans à deux ans, pour permettre une généralisation plus rapide. Le point étant fait sur les mesures prévues pour 2025, j’en viens à la question de l’avenir de la branche autonomie. À court et à moyen terme, les perspectives financières se détériorent. La dernière loi de financement de la sécurité sociale prévoyait un solde positif ou à l’équilibre jusqu’en 2027. Les nouvelles prévisions sont plus pessimistes : la branche serait déficitaire de 400 millions d’euros dès 2025 et à hauteur de 2,5 milliards d’euros à horizon 2028. En matière d’autonomie, le n’est pas envisageable. Je ne m’attarderai pas sur ce constat déjà bien connu de tous : dans le champ du grand âge comme dans celui du handicap, les besoins de financement sont massifs et incompressibles. Beaucoup d’établissements et services médico sociaux sont déjà en grande difficulté. Les départements aussi sont exsangues financièrement, et leur politique sociale en pâtit. À ce titre, nous ne pouvons que saluer les 200 millions d’euros que vous venez d’annoncer, monsieur le ministre, pour que la CNSA couvre mieux leurs dépenses d’APA et de PCH. Je rappelle par ailleurs que, dès 2030, c’est à dire dans cinq ans, la génération issue du baby boom passera la barre des 85 ans. Cela nous laisse très peu de temps pour répondre aux grands enjeux du virage domiciliaire, de la prévention et de l’attractivité des métiers. Aussi, comment s’organiser pour apporter ces réponses ? Le cœur du sujet réside dans le financement. Nous vous proposerons, dans le cadre de ce PLFSS, une première solution avec la mise en place d’une « contribution de solidarité par le travail de poser les jalons d’une réforme structurelle – pourquoi pas, monsieur le ministre, dans le cadre du projet de loi Grand Âge tant de fois promis ? Très bien ! Une partie de ces recettes pourrait aussi contribuer au remboursement des aides techniques destinées aux personnes en situation de handicap, mais il reviendra au Gouvernement de décider En définitive, mes chers collègues, si un effort est consenti dans le cadre de ce PLFSS, la question de l’avenir de la branche autonomie demeure entière. Très bien

la commission des finances a décidé à la majorité d’émettre un avis favorable sur ce texte, sous réserve des modifications qui seront apportées en séance. En effet, le présent Gouvernement hérite d’une situation dont il ne peut être tenu responsable. Il propose, de plus, des mesures de redressement significatives, qui s’appuient sur des hausses de recettes et des baisses de dépenses. Seront elles suffisantes ? Je ne le pense pas, malheureusement. Depuis 2020, la situation des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale s’était légèrement redressée, même si un déficit de près de 11 milliards d’euros demeurait en 2023.

Deux raisons expliquent cette aggravation. La première, c’est que les recettes seraient inférieures de 6,6 milliards d’euros aux prévisions, en raison d’hypothèses macroéconomiques trop optimistes, dont nous avons malheureusement l’habitude.

Un tel déficit est aussi lié à des hausses de dépenses non financées. Le Ségur de la santé représente ainsi un surcoût de près de 13 milliards d’euros par an.

l’année 2025, le Gouvernement anticipe un déficit de 16 milliards d’euros, inférieur de 2 milliards d’euros à celui de 2024. Il présente à cette fin des mesures intéressantes, tant des baisses des dépenses que des hausses des recettes.

Des hausses sont prévues notamment la refonte des allégements généraux de cotisations sociales – c’est une réforme intéressante, mais qui appelle des adaptations pour ne pas trop affecter l’emploi. Quant à l’augmentation prévue du taux de cotisation employeur de la CNRACL, elle pèsera très lourdement sur les comptes des collectivités territoriales, en contradiction avec la volonté du Gouvernement de réduire fortement les dépenses De plus, en raison du dispositif de compensation démographique, la CNRACL devrait verser près de 500 millions d’euros aux autres régimes de retraite en 2025. Est il bien normal de ponctionner un régime en déficit et de demander aux collectivités de cotiser davantage pour d’autres régimes ? régimes ? Je ne le crois pas. Un compromis plus acceptable pour les collectivités doit être trouvé sur ce sujet. La commission des affaires sociales propose une piste intéressante en ce sens. Les dépenses de la sécurité sociale ne devraient augmenter que de 2,8 % en 2025. Cet objectif est très volontariste, pour ne pas dire optimiste. Je note que des mesures d’économies sont proposées sur l’Ondam, pour un montant de 1,6 milliard d’euros. solde de la branche vieillesse devrait être contenu par rapport à 2024 grâce aux mesures de report de la revalorisation des retraites à hauteur de l’inflation. J’en viens au sujet que j’ai choisi d’approfondir en tant que rapporteur pour avis sur le PLFSS, à savoir le poids du système des retraites sur la dépense publique. En effet, dans la plupart des régimes de retraite, les cotisations ne sont pas suffisantes pour couvrir le niveau des pensions. En particulier, concernant les régimes de retraite des fonctionnaires publics, l’État augmente artificiellement chaque année les taux de cotisation employeur, afin de combler les déficits. Un même système est appliqué à la CNRACL. Si un taux de cotisation identique à celui du secteur privé était appliqué, le niveau des cotisations employeur serait beaucoup plus faible. Une présentation unifiée de ces éléments serait nécessaire, comme le recommande d’ailleurs notre collègue Sylvie Vermeillet… Notre excellente collègue ! … pour les retraites de la sphère publique.

Or la gestion à venir de la dette sociale interroge. En l’absence d’une nouvelle loi organique, aucune nouvelle reprise de dette par la Cades n’est possible. L’Acoss bénéficie de conditions d’emprunt moins avantageuses que la Cades, même en tenant compte des mesures du présent projet de loi.

Cela a été dit, l’Assemblée nationale n’est pas parvenue au terme de l’examen de ce texte dans le délai imparti. Par conséquent, notre chambre sera la seule en mesure de se prononcer en première lecture sur l’ensemble des mesures de ce PLFSS.

d’abord, nous ne souhaitons pas dégrader le solde proposé par le Gouvernement. Nous savons que nos partenaires scrutent la séquence budgétaire de notre pays et que la crédibilité de la France est en jeu, de même que celle des travaux du Sénat. Il convient donc de faire preuve de responsabilité.

En somme, à nos yeux, chacun doit participer, mais de façon équitable et, surtout, en préservant l’emploi et la qualité des services. Cette feuille de route se traduit par des choix forts, dont nous aurons l’occasion de débattre. Je veux revenir plus particulièrement sur trois d’entre concernant les allégements généraux, nous avons accepté le principe d’une maîtrise d’un dispositif dont le coût a augmenté de près de 20 milliards d’euros ces trois dernières années.

D’une part, je pense que nous partons sur des bases plus claires, voire plus sincères, que les années précédentes. D’autre part, le Sénat aura sans doute une influence beaucoup plus forte qu’à l’accoutumée sur la copie finale. Nous en prendrons la responsabilité.

Or c’est justement parce que nous sommes soucieux de ces principes que je défends devant vous cette exception d’irrecevabilité et vous demande donc de renvoyer le texte à l’Assemblée nationale.

La procédure retenue par le Gouvernement a abouti à enjamber purement et simplement l’Assemblée nationale. Elle n’est conforme ni à nos institutions, ni au parlementarisme, ni à l’exercice de la souveraineté nationale. Que s’est il passé à l’Assemblée nationale ? En commission, les deux premières parties du PLFSS ont été rejetées, ce qui, déjà, n’est pas banal. En séance publique, la deuxième partie, sur les recettes, a été adoptée

La raison, à l’inverse, c’est de sauver notre système de protection sociale en lui assurant des recettes supplémentaires, afin de le ramener progressivement à l’équilibre.

à l’Assemblée nationale. Aussi, le 5 novembre à minuit, alors que, de jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, il était possible de prolonger le débat tard dans la nuit – les députés y étaient prêts, du moins ceux de gauche

Y avait il une autre voie possible ? Bien sûr ! Celle de la coconstruction. Alors que le Premier ministre avait indiqué que le PLFSS était « perfectible »,

Le Gouvernement nous donne un rôle qui n’est pas le nôtre et qui n’est pas conforme à nos institutions. Ce rôle, nous n’en voulons pas. Nous n’avons aucune légitimité à nous substituer aux députés et à nous rendre complices d’un déni démocratique. Pensez vous vraiment que la démocratie se porte si bien, en France et partout ailleurs, que l’on puisse la maltraiter, la contourner, la nier ? Il nous semble, à l’inverse, que nous devons être exemplaires dans l’exercice démocratique, plus que jamais ! C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous invite à voter cette exception d’irrecevabilité.

Le scrutin est ouvert.

Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer l’exception

les conditions dans lesquelles nous entamons l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont particulièrement préoccupantes. En effet, le Gouvernement a détourné l’usage de l’article 47 1 de la Constitution pour empêcher l’examen du PLFSS pour 2025 à l’Assemblée nationale. Vous avez, dans un premier temps, choisi cette option parce que vous connaissez l’hostilité des Français à l’égard de l’utilisation de l’article 49.3, que vous affectionnez particulièrement.

ont rendu impossible l’examen de la totalité du PLFSS dans le délai imparti de vingt jours. Les rappels au règlement à répétition et les secondes délibérations sur les votes ont permis au Gouvernement, minoritaire, de transmettre au Sénat la version initiale du texte, les amendements qui lui convenaient. Il faut dire que l’examen du texte à l’Assemblée nationale a été une véritable déroute pour le Gouvernement, qui a accumulé les défaites et les défections dans son propre camp. Les députés de gauche avaient réussi à faire adopter près de 20 milliards d’euros de recettes nouvelles, notamment au travers d’un amendement visant à soumettre à cotisations sociales les dividendes, l’intéressement, la participation et les plus values de levée vente d’actions. Le Gouvernement a perdu sur les amendements portés par la gauche, mais aussi contre ses propres troupes. Ainsi, la suppression de l’article 6, qui prévoyait une toute petite réduction des cadeaux aux entreprises, a été votée par les députés du Rassemblement national, de la droite et du centre. Heureusement, le Gouvernement, sans majorité à l’Assemblée nationale, peut compter sur ses soutiens ici, au Sénat, pour faire le sale boulot. Il faut le dire aussi, les conditions sont réunies pour priver le Parlement d’un débat démocratique sur un budget de 662 milliards d’euros. Le PLFSS pour 2025 est un budget d’austérité, dont les deux tiers des économies reposent sur les assurés sociaux, avec une baisse de leurs prestations de retraites, une réduction des indemnités journalières, une hausse des franchises médicales et – dernière en date – une diminution du remboursement des médicaments. Ce texte austère se borne à prévoir les objectifs de dépenses des branches de la sécurité sociale, mais ne contient aucune mesure sur les sujets qui sont pourtant au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Ce PLFSS pour 2025 ne prévoit aucune mesure sur l’accès aux soins, rien sur la formation des professionnels de santé, rien sur les fermetures de services d’urgences, rien sur l’installation des médecins dans les déserts médicaux, rien sur le contrôle des crèches privées lucratives, rien sur la défense de la souveraineté de la France en matière de médicaments, rien sur la lutte contre les morts au travail

Vous ne pourrez pas utiliser l’argument des délais de préparation du PLFSS, alors que les services de Bercy travaillaient sur ce texte depuis le printemps dernier et que les mesures figurent dans le plan budgétaire et structurel de moyen terme (PSMT) transmis à Bruxelles.

Nous le savons et nous le vivons dans nos territoires, avec l’inflation et la pauvreté, le sujet de la santé fait partie des premières préoccupations des Français. Comme chaque année, notre groupe a donc décidé de déposer une motion tendant à opposer la question préalable pour marquer son opposition à la philosophie qui sous tend ce texte.

que vous en disiez, le Gouvernement poursuit et aggrave les politiques de réduction des dépenses de la sécurité sociale en 2025. S’agissant des dépenses de santé, le gouvernement prévoit une augmentation des dépenses de 2,8 %, soit, après la déduction du taux d’inflation, une hausse de 1,8 %. Si l’on retranche la hausse des cotisations de la CNRACL, la hausse des dépenses de santé sera de seulement 0,6 % en 2025. Le budget de l’assurance maladie progresse, donc, mais, si on le compare aux besoins existants, nous sommes à des années lumière de ce qu’il faudrait investir.

Le Gouvernement refuse d’entendre la souffrance des personnels des secteurs de la santé et du médico social, ainsi que celle des patientes et des patients qui n’ont plus de médecin traitant, que ce soit en zone urbaine ou, pis encore, en zone rurale. Six millions de nos concitoyens sont concernés par cette triste réalité. Ils attendent des heures sur les brancards dans les couloirs des hôpitaux, faute de moyens et de personnels dans ces

Ne faudrait il pas tirer le signal d’alarme lorsque l’on constate que 42 % des maternités ont fermé depuis 1995 sur notre territoire ? Le Gouvernement reste sourd aux revendications des organisations syndicales pour améliorer l’attractivité des métiers et les niveaux de rémunération, alors même que les hôpitaux sont au bord de l’implosion et que la médecine de ville est à bout de souffle : 85 % du territoire français est un désert médical et 66 % des Ehpad

de cotisations patronales, ou même qu’on les conditionne, par exemple, au maintien dans l’emploi en France ou au respect de l’environnement. En 2023, les exonérations de cotisations représentaient 16 % des 486 milliards d’euros d’excédents bruts des entreprises. La part des contributions des employeurs dans le financement du régime général est passée de 72 % en 1980 à 50 % en 2000, pour atteindre 28 % en 2022. Pour la branche maladie, la contribution des employeurs ne représente plus que

les assurés sociaux cotisent toujours plus longtemps, devront payer plus cher leurs complémentaires santé, financeront la sécurité sociale à la place des entreprises en faisant leurs courses la TVA seront moins bien remboursés en cas d’arrêt maladie ou lors de leur rendez vous chez le médecin. Ce PLFSS est donc particulièrement injuste, puisque les trois quarts des efforts reposent sur les assurés sociaux, sans que soient augmentées les cotisations des entreprises,

de loi est loin des attentes des Français. Il fait payer aux plus fragiles le déficit, alors que d’autres recettes sont possibles – nous sommes d’accord sur ce point avec Mme la rapporteure générale. Ce texte comptable est loin de la justice sociale que nous défendons. Pour ces raisons, nous voterons en faveur de la motion

la parodie de démocratie qui consiste à n’examiner que vos seuls amendements, qui tendent à modifier le niveau de l’effort d’austérité imposé aux hôpitaux, aux collectivités et aux citoyens, sans jamais remettre en cause le principe même de l’austérité. Le Gouvernement a interprété de manière extensive l’article 47 1 de la Constitution, afin de gagner la course contre la montre, faute de disposer d’une majorité à l’Assemblée nationale. En déposant plus de 1 300 amendements, les députés du bloc de la majorité ont impossible l’examen du PLFSS dans les délais constitutionnels. Selon vos dires, il s’agit des règles du débat démocratique. Pourtant, souvenez vous

Le scrutin est ouvert.

contrat social qui nous engage collectivement. Il incarne notre devoir de garantir l’équité médico sociale sur l’ensemble de nos territoires, notamment outre mer, conformément aux principes les plus fondamentaux de notre République. nous devons aussi améliorer la fluidité entre la sécurité sociale et les complémentaires santé, tant pour lutter plus efficacement contre la fraude que pour mieux cibler les besoins de prévention, qui demeurent le parent pauvre de notre système de santé. santé. En responsabilité, nous devons surmonter les carcans parfois hypocrites de nos appartenances politiques, pour prendre les décisions nécessaires et justes pour l’avenir de notre pays, de nos enfants et des Français. La parole

Tous nous ont permis d’entamer ces débats dans la clarté, alors que la tâche n’était pas si simple. En effet, mardi 5 novembre à minuit, l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025

Ainsi, comme l’a évoqué le rapporteur pour avis de la commission des finances Vincent Delahaye, le déficit de la sécurité sociale se dégrade de nouveau en 2024. Il atteint 18 milliards d’euros, soit 7,5 milliards d’euros de plus que la prévision mentionnée dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce dérapage provient très majoritairement de recettes inférieures aux prévisions.

fait peser un risque réel sur la pérennité du système obligatoire et universel pensé par le Conseil national de la Résistance et créé par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945.

les baisses de cotisations patronales ne sont pas toujours efficaces sur l’emploi et le niveau des salaires, alors qu’elles dégradent substantiellement les comptes sociaux. Les exonérations de cotisations sociales dont bénéficient les employeurs affiliés au régime général atteignaient 50 milliards d’euros en 2019. Elles ont ensuite connu une hausse spectaculaire de de 13,1 % en 2022, avec un montant de 73,6 milliards d’euros, pour enfin se stabiliser à 75 milliards d’euros aujourd’hui. Par ailleurs, cette dynamique s’inscrit de plus en plus dans une généralisation des dispositifs d’allégement, qui ne sont plus autant ciblés sur des territoires, des secteurs particuliers ou de petites entreprises. Les aides publiques sont donc bien moins conditionnées au respect de critères de justice sociale et territoriale, alors que les besoins sont très clairement là.

Néanmoins, la mesure nous semble incomplète, puisqu’aucun dispositif de différenciation selon la nature de l’entreprise n’est prévu à ce stade. Il est pourtant injuste qu’un artisan plombier ou coiffeur soit logé à la même enseigne que des géants de la grande distribution ou des compagnies pétrolières.

La commission des affaires sociales du Sénat s’est prononcée en faveur d’un étalement sur quatre ans de la hausse des cotisations, ce qui nous paraît plus sage. Toutefois, le groupe RDSE reste très réservé au sujet de cette augmentation, qui, à titre d’exemple, représenterait pour la ville de Mende, dans le département de la Lozère, une charge supplémentaire de 136 000 euros.

Comme à l’accoutumée, notre groupe aborde cette période budgétaire de manière constructive. Pour cette raison, nous sommes par exemple satisfaits des mesures en faveur de la lutte contre les pénuries de produits de santé qui se manifestent ponctuellement dans nos pharmacies. Nous saluons également les financements supplémentaires pour le secteur de la santé mentale, en particulier des jeunes, et les moyens accrus pour les soins psychiatriques et psychologiques. d’un combat important, que notre groupe avait porté l’an dernier en compagnie de notre ancienne collègue, désormais ministre, Nathalie Delattre, au moyen d’une proposition de résolution invitant le Gouvernement à ériger la santé mentale des jeunes en grande cause nationale.

Pour conclure, vous l’aurez compris, nous défendrons nos amendements dans un esprit de responsabilité et nous nous prononcerons sur les propositions de nos collègues au cours des prochains jours,

dans un contexte politique difficile et face à une situation financière préoccupante pour l’État, la sécurité sociale affiche en 2024 un déficit de 18 milliards d’euros.

Ce constat, bien qu’il soit lourd, n’appelle ni à la fatalité ni à la résignation. Il doit au contraire nous pousser à une réflexion lucide sur nos réussites et nos erreurs, afin de nous inciter Parce qu’il résulte de causes que nous connaissons bien, ce déficit nous alerte sur les défis sociaux et financiers que nous devons relever. Le vieillissement de la population est une réalité démographique la baisse de la natalité en est une autre. Les dépenses de santé et de retraite augmentent, alors que les recettes tirées de la croissance, censées les accompagner, sont en berne. Ne nous trompons pas le déséquilibre des comptes de la sécurité sociale n’est pas conjoncturel. Les crises ont certes pesé, mais l’absence de réformes structurelles demeure la principale menace pesant sur notre système. ne résoudrons donc pas le problème en transférant les remboursements vers les mutuelles et les complémentaires santé. Le remboursement croisé des prestations

J’ai souvent dénoncé les actes médicaux redondants et autres examens inutiles, qui pèsent lourdement sur nos comptes et qui Je répète ce qui, loin d’être un simple discours de principe, est un fait admis par tous, notamment par nombre de professionnels de santé eux mêmes : l’inscription dans le dossier médical partagé de tous les actes médicaux doit devenir obligatoire

Nous devons encourager le parcours de soins et tisser les partenariats et le maillage nécessaires avec les autres professionnels de santé : c’est la clé de l’accès aux soins pour tous.

le déficit est persistant. C’est le signe qu’il faut repenser fondamentalement le système. Les trois régimes par répartition, privé, public et libéral, doivent être traités séparément, pour que chacun retrouve ou maintienne l’équilibre.

Pour augmenter les salaires et la compétitivité des entreprises, il faut trouver des ressources nouvelles sans pénaliser le travail et la productivité. Le groupe Union Centriste propose ainsi d’augmenter la TVA d’un point, à des biens de première nécessité, pour que les consommateurs partagent l’effort de justice sociale. En conclusion, si nous voulons ne pas laisser

avons à l’esprit les soignants et celles et ceux qui exercent les métiers du lien, victimes de conditions de travail de plus en plus difficiles et de rémunérations qui leur font tourner le dos à leur vocation, la mort dans l’âme. avons à l’esprit les gestionnaires d’établissements publics de santé, du secteur social ou médico social, qui, malgré leur travail rigoureux, ne parviennent plus à résorber des déficits devenus structurels.

Pis, il aggravera encore toutes ces situations, sans même réduire un déficit annoncé à 16 milliards d’euros. En effet, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Plutôt qu’aller chercher de nouvelles ressources pour financer notre système de protection sociale, en faisant par exemple contribuer les revenus financiers, qui échappent pratiquement à toute contribution à la solidarité nationale, plutôt qu’examiner sérieusement les exonérations de cotisations et les niches sociales qui grèvent de plus en plus et de plus en plus rapidement nos finances publiques, plutôt que responsabiliser l’industrie pharmaceutique, dont les choix stratégiques sont davantage guidés par le taux de rentabilité que par la santé collective, vous souhaitez faire reposer presque exclusivement les efforts sur nos concitoyens. Vous vouliez économiser 3,6 milliards d’euros grâce aux retraites en reportant de six mois l’indexation des pensions sur l’inflation. Face au mécontentement, vous êtes contraints de reculer, mais 56 % des retraités seront privés de l’entièreté de la revalorisation attendue, conduisant 9,5 millions d’entre eux à perdre du pouvoir d’achat. Plus encore

difficile de parler de solidarité quand les salariés sont ainsi mis à contribution, alors que la moindre diminution des exonérations de cotisations sociales est battue en brèche ! Quelque 4 milliards d’euros de moins sur les près de 80 milliards d’euros Plus globalement, qui peut raisonnablement penser qu’un objectif de dépenses de santé en augmentation de 2,8 % en 2025 est réellement tenable ? La Commission européenne y croit peut être, mais pas nos concitoyens,

Ce régime ne peut qu’amplifier un phénomène que nous ne connaissons déjà que trop bien : des hôpitaux exsangues, des agents usés, malgré leur dévouement, par des conditions de travail toujours plus difficiles…

une idée désormais majoritaire dans notre pays, même s’il y a débat – c’est légitime – sur l’endroit où il convient de placer le curseur de cette régulation. Ce PLFSS devrait en l’état être l’occasion d’établir un plan pluriannuel de financement du grand âge. Or, non seulement

le biais de motions adoptées en conseil d’administration, de nombreux Ehpad nous ont pourtant avertis de leurs difficultés à faire face à l’inflation de ces derniers mois et à l’insuffisante compensation des mesures de revalorisation salariale.

Un an et quatre ministres de la santé plus tard, force est de constater qu’il n’y a plus de capitaine pour orienter les finances sociales. Le budget 2024 de la sécurité sociale était manifestement insincère : le Gouvernement avait surestimé les recettes de près de 5 milliards d’euros

entre retraités et actifs, entre malades, supposément fraudeurs et profiteurs, et cotisants, entre travail et travailleurs. Après ces attaques contre « la sociale », la droite a eu la bonne idée de créer les lois de financement de la sécurité sociale. Chaque année, le Parlement examine désormais, à la place des travailleuses et des travailleurs, les comptes de la « sécu », pour constater les déficits successifs et pour réduire les droits sociaux, sans aucun cadrage pluriannuel de surcroît. planifier sur un an est déjà trop peu pour gouverner, une telle échéance n’a aucun sens si l’on veut garantir le fonctionnement de l’hôpital, nos retraites et nos prestations sociales. Cette année encore, le PLFSS présente un déficit : 18 milliards d’euros cette fois

nouvelle journée de solidarité déguisée, autrement dit, d’une nouvelle corvée d’Ancien Régime ! Nous nous opposerons à ces mesures. Toutefois, nous reconnaissons que tout n’est pas à jeter dans ce projet. Premièrement,

? Le texte reste plus qu’alarmant sur ce sujet, laissant aux mutuelles le soin de payer presque la moitié de ensemble est inquiétant. Plutôt que de restreindre les droits sociaux et faire payer les malades, donc les plus fragiles d’entre nous, vous auriez pu choisir d’autres mesures pour rétablir l’équilibre financier de la sécurité sociale. C’est ce que nous souhaitons défendre aujourd’hui.

en récupérant le manque à gagner des exonérations de cotisations non compensées. Ensuite, nous proposons de faire entrer la sécurité sociale dans le nouveau régime climatique, en mettant à contribution les responsables du changement du climat et de l’effondrement de la biodiversité, ainsi que les empoisonneurs, grâce à une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières.

Enfin, nous proposons de mettre en place une réelle fiscalité comportementale. L’idée n’est pas neuve : en 1861, le chansonnier Gustave Nadaud appelait déjà à « frappe[r] le vin et la bière » et à « n’épargne[r] point les tabacs

et que, cette fois, madame la ministre, notre vote sera respecté. En dernier lieu, nous souhaitons nous attaquer aux pratiques « anti santé publique » des industriels de l’agroalimentaire, en taxant les sucres ajoutés et les produits n’affichant pas le Nutriscore. Je compte sur vous,

La loi Grand Âge, madame la ministre, n’est toujours pas présentée : quand arrivera t elle ? Là encore, je compte sur vous. Vous l’aurez compris, face aux attaques à pas feutrés du « socle commun » contre les conquis sociaux, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires défendra le patrimoine de celles et de ceux qui n’en ont pas.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2025, tel qu’il est proposé par le Gouvernement, nous inquiète comme jamais, car il met à mal les fondements mêmes de notre protection sociale.

ni de résoudre les déficits ni de proposer la moindre trajectoire de retour à l’équilibre. Il vise à augmenter timidement les recettes et à réduire drastiquement les dépenses en les mettant à la charge des malades. Ce budget cache en réalité une vision politique que nous refusons : laisser filer les déficits pour simuler l’inefficacité de notre système de sécurité sociale, issu du Conseil national de la Résistance. En effet, nous nous éloignons toujours plus du principe selon lequel chacun participe selon ses moyens et bénéficie

des mutuelles ou des assurances privées conduit à les rendre inabordables pour les plus fragiles et à rompre le principe d’égalité d’accès aux soins. Je m’étonne que Les Républicains et la droite sénatoriale se soient associés à ce projet de budget macroniste, que nous pouvons qualifier d’insincère et d’infidèle par rapport aux principes que nous défendons. Mme la rapporteure générale exprime son attachement à notre sécurité sociale, elle aura l’occasion de soutenir certaines de nos propositions, nous laissant entrevoir quelques avancées au Sénat…

donnez ainsi le coup de grâce aux villes et aux départements, déjà exsangues. Pour pérenniser le système français, il est de notre responsabilité – c’est une exigence – d’assurer l’équilibre budgétaire des différentes branches de la sécurité sociale, lesquelles ne peuvent fonctionner avec un déficit permanent. Le peu de recettes nouvelles présentées ne permettra pas le retour à cet équilibre. Je reste étonnée de voir la majorité sénatoriale soutenir cette fuite en avant des déficits, alors que, dans ses rangs, on dénonce cette logique depuis des années. Nous avions perçu un signe positif avec la proposition faite par le gouvernement Barnier de réduire les insensés allégements généraux de cotisations. Nous proposons d’aller plus loin avec une sortie des exonérations des salaires excédant deux Smic. Ainsi, nous dégagerons 8 milliards d’euros de recettes sur les 80 milliards d’euros d’allégements généraux. Nous irons chercher les exonérations ayant montré leur inefficacité inefficacité pour l’emploi et pour la compétitivité de nos entreprises. Nous compléterons ces ressources par une contribution des revenus exceptionnellement élevés et par une fiscalité comportementale chère à notre rapporteure générale. Toutefois, d’autres recettes proposées par Mme le rapporteur Deseyne pour la branche autonomie nous excèdent. travailler les seuls salariés un jour de plus sans être payés n’est respectueux ni de la justice sociale ni du travail. Notre groupe propose des recettes raisonnables, à la juste hauteur des besoins, pour assurer un retour à l’équilibre à terme, sans ponctionner toujours plus les salariés, les malades ou les retraités. Annonce du report de la revalorisation

Côté dépenses, nous nous opposerons à toute augmentation du reste à charge qui pèse sur les malades et sur les plus vulnérables. Je pense à la hausse du ticket modérateur ou à la diminution des indemnités journalières. Nous revendiquons une loi de programmation pluriannuelle pour la santé, tout comme une loi pour le grand âge, promise, mais toujours pas présentée

à la hauteur des enjeux. Invisibilisée dans votre budget, la santé mentale est pourtant supposée être la grande cause du Premier ministre. Invisibilisée, la politique familiale l’est aussi alors que les familles monoparentales attendent des dispositifs nouveaux, notamment la réforme du congé parental. Invisibilisés, le renoncement aux soins et les prises en charge tardives faute de médecins le sont également. Nous, socialistes, considérons qu’il est possible de concilier la justice, fiscale et sociale, et le rétablissement des comptes de la sécurité sociale. Nous nous battrons pour préserver l’accès aux services publics et aux soins, de la crèche à l’Ehpad. Nous refuserons de vendre la protection sociale à des acteurs ayant une logique lucrative, dont les effets délétères sont dévoilés par de nombreux scandales. J’espère que le Gouvernement et sa majorité sénatoriale se saisiront du sérieux de nos propositions et que nous sortirons de notre débat avec un budget structurant,

la France fit le choix historique de confier à la Nation et au Parlement le financement et la prise en charge de la solidarité nationale, des politiques de santé et des risques de la vie. D’autres pays n’ont pas fait ce choix et ont laissé au privé la gestion de la santé des populations, source parfois d’efficacité et de rigueur comptable, très souvent d’un lot d’inégalités et d’exclusions. politiques sont des dépenses, mais des dépenses supposées utiles, solidaires et justes, qui permettent à nos concitoyens d’être pris en charge de la meilleure des façons et de la plus égale des manières, partout où ils se trouvent. mes chers collègues, la justice n’exclut pas la responsabilité. La dette sociale participe à part entière de la dette de l’État. Sous le septennat douloureux du président Macron, cette dette a continué à se creuser malgré les réformes injustes, particulièrement celle des retraites qui, sans être une trahison, puisqu’elle fut largement assumée avant la réélection du président, n’en a pas moins été un acte de brutalité sociale envers les travailleurs les plus modestes. Comme chaque année, le même questionnement lancinant nous saisit. Quelque 662 milliards d’euros de dépenses de sécurité sociale, près d’un quart de notre richesse nationale, et une progression prévue de 18 milliards d’euros : normalement, mes chers collègues, avec une telle somme, nos hôpitaux devraient être les meilleurs du monde, notre espérance de vie progresser notre natalité être dynamique ; les Français devraient pouvoir se soigner sans crainte de la facture, de l’attente d’un spécialiste ou de la file dans un service d’urgence, et sans s’inquiéter d’obtenir le médicament nécessaire. Pourtant, partout où nous portons nos regards, la situation est dramatique. Nos soignants souffrent encore et toujours. Les proches aidants, soutien vital à notre système de santé, permettent, par leur abnégation, d’économiser des centaines de milliards d’euros et apportent à des millions de nos concitoyens les soins et l’attention nécessaire pour mener la vie la plus normale le plus longtemps possible. Plus grave encore, notre natalité, ciment de la prospérité et, soit dit en passant, de tout l’équilibre financier de notre système social, est en baisse structurelle. Dans de nombreux territoires, même les plus urbanisés, le manque de médecins se conjugue maintenant avec le manque de médicaments, voire avec le manque de pharmacies. Mes chers collègues, le constat est sombre, mais il est malheureusement juste. La question n’est pas tant de savoir si nous dépensons trop, mais surtout pourquoi aucun paramètre social et sanitaire ne s’améliore. Dans une fuite en avant austéritaire et à l’effet récessif, le Gouvernement souhaite rogner les droits sociaux des Français. Si des économies sont nécessaires, elles ne doivent ni toucher aux classes populaires et moyennes, ni toucher à la France laborieuse, ni diminuer les droits sociaux des Français, alors même que la récession revient.

Face à ce constat, il n’y aurait qu’une solution pour préserver notre système social : la rupture. La rupture avec des politiques nocives, la rupture pour améliorer le coût du travail, la rupture pour organiser un système de retraites plus juste, incitant à commencer le travail le plus tôt possible et non à connaître la pénibilité la plus longue qui soit, la rupture pour faire bénéficier prioritairement les Français des fruits sociaux des lourds impôts dont ils s’acquittent par leur travail. ils s’acquittent par leur travail. La rupture, nous craignons que vous n’y soyez favorables. Je disais déjà au début du mois d’octobre dernier que le problème de la classe politique française était non pas sa compétence, mais son conformisme. Dès lors, si rupture il doit y avoir, avant d’être financière, elle doit être politique. Montrez

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres,

Le PLFSS qui nous est proposé s’intègre dans le plan du Premier ministre, lequel souhaite ramener le déficit de 6,1 % à 5 % du PIB en 2025. Il vise à limiter le déficit de la sécurité sociale à 16 milliards

Il n’est pas question d’une diminution des soins pour nos compatriotes. Tout d’abord, 4 milliards d’euros d’économies proviendront de la diminution des allégements de cotisations patronales. Je suis d’accord avec la proposition de la rapporteure, qui souhaite protéger les allégements proches du Smic.

sont envisagés la modération des dépenses de santé avec la hausse du ticket modérateur – il faudra en tenir compte pour les Français qui n’ont pas de mutuelle – et un meilleur encadrement des dépenses de certains examens complémentaires.

le non retour à la consultation, ce qui signifie souvent l’arrêt du traitement. Je souhaite exprimer mon accord avec les propositions des rapporteurs des différentes branches : lutter plus intensément contre la fraude avec une carte Vitale sécurisée, favoriser la vaccination contre les papillomavirus et les méningocoques et la prévention, lutter contre les actes redondants et favoriser l’utilisation du dossier médical partagé (DMP), contrôler l’utilisation des dispositifs, lutter contre la pénurie de médicaments, renforcer la prévention au travail et la lutte contre l’usure professionnelle, enfin, prendre en compte la dénatalité.

en effet issus de familles modestes. Nous espérons que la réduction du seuil d’exonération des cotisations sociales pour les apprentis au 1janvier 2005 n’aura pas d’effet négatif. Nous devons aussi redonner sa valeur au travail. À

pour les parlementaires : ils sont prisonniers d’un texte, sous la menace des canons Caesar de l’article 40 ou des tirs de HK 416 de l’article 45

la covid 19 fut un révélateur. Cette désintégration s’explique par des maux structurels et plusieurs décennies de renoncement. Le système de santé français est fondé sur les principes d’universalité, d’égalité, d’accessibilité et de qualité. Alors qu’il a longtemps figuré parmi les plus performants, il est aujourd’hui en cours d’effondrement. Nous ressentons tous le besoin d’une réforme structurelle, mais elle ne peut venir d’un PLFSS trop restreint, sans vision d’avenir, annuel et désormais stérile, tant il est tendu vers le respect du dogme de la gratuité de tout pour tous et

Le gouvernement actuel est trop récent pour que l’on puisse lui imputer la responsabilité intégrale de ce PLFSS, mais il doit pouvoir, dans les mois à venir, se débarrasser du carcan purement financier qui pèse sur la santé. Le sauvetage de notre système de santé passe par une profonde transformation, vous l’avez dit, madame la ministre. Le premier principe hérité de 1945 est l’universalité : tous nos concitoyens jouissent des mêmes droits fondamentaux du fait de leur humanité.

À quand une loi de programmation structurelle sur l’organisation et le financement de la santé qui donnerait une visibilité à long terme à l’ensemble des acteurs de santé sur notre territoire ?

À quand un investissement significatif dans la prévention, à partir des données de santé dont nous disposons et qui sont, me semble t il, particulièrement nombreuses, de qualité et complètes ?

Le troisième principe est l’accessibilité. On entend souvent dire que les hôpitaux ont reçu beaucoup d’argent ces dernières années. Les personnels ont certes bénéficié de revalorisations salariales, mais les établissements n’ont pas vu leurs effectifs augmenter Circonstance aggravante, les crédits accordés pour financer ces augmentations n’ont pas été entièrement alloués, en raison du déficit de la sécurité sociale. Face aux critiques sur la dégradation des conditions de travail liée au manque de personnel, le message affiché est de ne pas toucher à l’emploi. La variable d’ajustement consiste à geler des emplois par des différés de recrutement et à réduire les dotations aux investissements, ce qui est grave pour l’avenir de l’hôpital. Aussi, face au manque de personnel, on ferme des lits. Ne pourrait on pas prendre le temps d’analyser et d’agir autrement, en instaurant, par exemple, un moratoire d’une année de non fermeture de lits d’hôpitaux ?

Le maintien en bonne santé de nos concitoyens grâce à une diffusion des mesures de prévention dans tous les domaines, y compris dans celui de la nutrition, est nécessaire, même si l’on doit mettre en place des mesures de rétorsion, mal comprises par quelques uns.

La prévention doit prendre une place centrale dans tout système de santé. Le vieillissement est une chance, mais il peut devenir une menace s’il ne se fait pas en bonne santé. Faisons de la sécurité sociale une institution démocratique, gérée par des représentants des usagers. Gérons la santé de nos concitoyens en prenant en compte leurs besoins et leur lieu de vie. Et faisons confiance aux professionnels de santé.

qui est marqué par un effort inédit en faveur du redressement des finances publiques et des comptes sociaux. La pandémie de covid 19 et les crises sociale et économique qui lui ont succédé ont en effet entraîné une augmentation importante des dépenses de l’ensemble des administrations publiques. Face au déficit de 18 milliards d’euros des comptes de la sécurité sociale pour l’année 2024 et aux perspectives négatives pour les quatre années à venir, il nous revient d’engager des efforts importants pour reprendre la maîtrise de nos comptes sociaux et ne pas laisser aux générations futures une dette qui serait insoutenable. qui serait insoutenable. Cela étant, le PLFSS pour 2025 prévoit un budget de 662 milliards d’euros pour la protection de nos concitoyens, soit la moitié de la dépense publique et le tiers de notre richesse nationale.

Contrairement à ce que certains affirment, ce PLFSS est donc un budget non pas d’austérité, mais de responsabilité. Le groupe RDPI soutient résolument la trajectoire de réduction des déficits publics voulue par le Premier ministre et son gouvernement. Si le déficit actuel et prévisionnel des comptes sociaux invite à mener des réformes structurelles et à accroître l’efficience de notre système de santé, nous considérons avec prudence toute mesure qui viendrait affecter les politiques de soutien à l’emploi que nous avons menées avec succès depuis sept ans.

Cette exigence en faveur de l’emploi, notamment des bas salaires, nous l’aurons également concernant les apprentis et les jeunes entreprises innovantes.

L’autonomie des personnes âgées et handicapées constitue une autre priorité pour notre groupe. Dans un contexte budgétaire très contraint, nous apprécions l’effort budgétaire proposé en faveur de la cinquième branche. Il nous faudra toutefois faire plus pour nos Ehpad. Le récent rapport sénatorial sur la situation de ces établissements, dont j’ai été corapporteure, démontre l’urgence de financer davantage ce secteur et contient des solutions que j’invite le Gouvernement à reprendre dans les prochains mois.

Le groupe RDPI, composé pour moitié de sénateurs ultramarins, y veillera. Vous l’aurez compris, nous soutiendrons de manière exigeante ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, que nous chercherons toutefois à améliorer, afin de mieux protéger nos concitoyens, tout en garantissant à terme la soutenabilité de notre système de protection sociale. La parole

le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, que nous examinons aujourd’hui, répond certes aux impératifs budgétaires immédiats, lesquels doivent nous obliger à penser des réformes systémiques essentielles au maintien de notre protection sociale. force est de constater que les simples ajustements qui devraient garantir la pérennité et la soutenabilité de notre système de solidarité demeurent, et demeureront, insuffisants. Il faudra s’interroger sur les dépenses parfois surprenantes et excessives.

Parmi les mesures phares de ce PLFSS, on relève un effort notable de 1,2 milliard d’euros pour le secteur médico social, afin notamment de renforcer l’attractivité des métiers de l’aide à domicile, en revalorisant les conditions de travail et en encourageant la montée en charge des mesures récentes, telles que la tarification des soins infirmiers Le budget alloué à l’aide à domicile inclut également une subvention exceptionnelle de 100 millions d’euros aux départements. Il s’agit de renforcer la mobilité et le soutien des personnels du secteur. Une nouvelle fois, ce montant est en deçà des attentes des départements, qui connaissent de grandes difficultés financières.

Le recrutement de 6 500 professionnels en Ehpad, soutenu par un financement de 380 millions d’euros, constitue aussi un pas en avant. Cependant, je veux ici que nous nous interrogions sur la notion d’attractivité, devenue trop habituelle, voire automatique. Nous ne connaissons pas un seul secteur d’activité qui ne connaisse pas un déficit de recrutement… Les conditions salariales et l’accès à des formations sont évidemment une partie de la réponse. Le Ségur de la santé y avait déjà partiellement répondu.

Le lancement d’une campagne de promotion dans le secteur médico social est une initiative bienvenue, sur le modèle de ce que font nos armées, pour valoriser ces métiers tournés vers l’autre. tournés vers l’autre. L’effort consenti pour financer le déploiement de 50 000 solutions d’accueil pour les personnes en situation de handicap mérite d’être relevé. Nous savons qu’une telle offre est indispensable pour assurer un accompagnement digne et adapté à chacun et pour soulager les familles, qui portent souvent seules cette charge. À cet égard, je me réjouis tout particulièrement de constater que nous faisons justement un pas de plus pour les proches aidants, dont le rôle est aussi essentiel qu’épuisant. Ce soutien va dans le sens de la stratégie nationale 2023 2027, qui prévoit des solutions de répit pour ces aidants, afin de leur permettre de souffler et de retrouver des forces pour accompagner au mieux leurs proches. Cependant, je tiens à souligner que le congé de proche aidant n’est toujours pas adapté pour être pleinement effectif. Mes chers collègues, je veux ici vous alerter collectivement sur le financement global de notre système de sécurité sociale. Vous le savez, l’augmentation de 63 milliards d’euros de nous impose aujourd’hui une gestion responsable et rigoureuse. La crise sanitaire a nécessité des financements d’urgence, que personne ici ne remet en cause, mais il est temps de revenir à un cadre de dépenses plus équilibré, pour garantir la pérennité de notre système. Aussi, dans ce contexte de nécessaire rigueur budgétaire, il est crucial de réfléchir à des sources de financement complémentaires, pour répondre aux besoins spécifiques de notre système de solidarité, en particulier pour la prise en charge de l’autonomie. Le temps est non pas à de nouvelles dépenses, mais à la sobriété. J’aurais pourtant voulu vous parler de prévention et ouvrir la réflexion sur l’abaissement à 45 ans de l’âge d’éligibilité aux dépistages de

En complément de la première journée de solidarité instaurée en 2004, cette contribution permettra d’augmenter les ressources de la branche autonomie de près de 2,5 milliards d’euros. Il s’agit d’un soutien essentiel pour aider les 86 % des Ehpad qui sont en grande difficulté et menacent de fermer, ou encore pour financer le remboursement intégral des fauteuils roulants. Surtout, à quand une véritable réforme de notre système de santé ? J’ai l’impression que, chaque année, nous faisons les mêmes constats et nous contentons de simples aménagements à la marge…

de vous faire une proposition, monsieur le ministre, que vous pourriez reprendre à votre compte, concernant le remboursement des équipements de santé en matière optique et auditive. Face à l’évolution des usages vers une logique plus consumériste et à l’augmentation continue des dépenses, un ajustement des règles de remboursement pourrait se révéler pertinent envisager un allongement de la périodicité de remboursement de deux à trois ans. En conclusion, le groupe Union Centriste votera ce texte, tout en appelant de ses vœux des réformes courageuses et des solutions durables pour garantir la pérennité de notre modèle de protection sociale. La parole

est à M. Bernard Jomier. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, depuis deux ans, alors que les coûts liés à la pandémie se sont estompés, la majorité sénatoriale n’a pas eu de mots assez durs pour dénoncer la trajectoire de déficit des comptes de la sécurité sociale. Et elle avait raison ! Mais voilà, parvenue au gouvernement, cette même majorité nous annonce 60 milliards d’euros de déficit en quatre ans et ne réduit nullement le déficit cette année. Quelle déception ! chers collègues de la majorité sénatoriale, ayez au moins celle de l’action. Il est possible, il est raisonnable, il est nécessaire de ramener la sécurité sociale à l’équilibre en trois ans, comme l’a indiqué Annie Le Houerou.

les aliments ultratransformés. Vous avez ouvert ce dossier. Certains dans cet hémicycle proposent d’infliger deux points de hausse de TVA à tous les Français. Pour notre part, nous

des taux de rentabilité à deux chiffres et où les actes se multiplient, déconnectés des besoins de santé, quand par ailleurs trop de nos concitoyens n’accèdent plus aux soins nécessaires. La gabegie est insupportable en temps de pénurie. Nous proposons une gestion responsable et solidaire,

nous ne voulons pas seulement bien gérer la sécurité sociale : nous voulons transformer en profondeur l’élaboration du budget santé du pays. Nous proposons d’en renverser la logique actuelle, qui est centralisée, court termiste et déconnectée de la délibération sur les besoins de santé et les priorités de santé publique. Jamais notre pays ne mènera l’indispensable virage de la prévention dans le cadre actuel. Il faut changer la loi, pour que le travail collectif sur le budget de la santé commence chaque printemps dans les départements, sous le double pilotage des agences régionales de santé et des élus, avec la participation de l’ensemble des acteurs de santé et des usagers.

La promesse de tout changer après la pandémie s’est évanouie. Vous ne changez rien, promettant toujours pour demain, ce qui ne vous engage à rien, alors que notre sécurité sociale mérite d’être mieux gérée que ne l’est l’État. La parole

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, notre modèle social, qui fait la fierté de notre pays, est aujourd’hui confronté à une situation critique. Le déficit des finances sociales, anticipé à 18 milliards d’euros pour 2024, dépasse largement les prévisions initiales. Si nous ne réagissons pas rapidement, ce montant pourrait atteindre 28 milliards d’euros dès 2025. Il est de notre responsabilité collective de préserver et de renforcer ce pilier fondamental de notre société, car, derrière ces chiffres, c’est l’avenir de notre système de santé qui est en jeu. Ce défi est une chance de transformation, une occasion de redéfinir ensemble un équilibre qui concilie la soutenabilité financière et les attentes des Français. Notre ambition doit être claire : construire un système de santé plus efficace, plus accessible et surtout capable de répondre aux besoins futurs. En investissant dans la prévention, nous pouvons non seulement protéger la santé de nos concitoyens, mais également réduire les coûts pour notre système de soins. La vaccination, par exemple, est un outil puissant elle sauve des vies, prévient des maladies graves, réduit les hospitalisations et se révèle économiquement judicieuse. Nous devons aller encore plus loin en matière de politique vaccinale. Je proposerai un amendement visant à intégrer la promotion de la vaccination dans les rendez vous de prévention. ailleurs, une politique de vaccination locale, renforcée et mieux coordonnée avec les agences régionales de santé permettrait d’améliorer l’accès aux vaccins sur tout le territoire, y compris dans les zones les plus isolées. Les défis auxquels nous faisons face appellent également des solutions audacieuses et innovantes. La fiscalité comportementale en est une : en dissuadant la consommation de produits nocifs comme le tabac ou les boissons sucrées, nous protégeons nos concitoyens tout en réalisant des économies substantielles. Une hausse progressive du prix du tabac, par exemple, pourrait sauver des milliers de vies, tout en réduisant la charge financière liée aux maladies qu’il provoque. Ce n’est pas une utopie : des initiatives passées, comme le plan Cancer ou les hausses fiscales décidées de 2017 à 2020, ont démontré leur efficacité. Réduire le nombre de fumeurs, c’est diminuer le nombre de maladies chroniques, les hospitalisations et les coûts pour la sécurité sociale. C’est investir pour des Français en meilleure santé. Enfin, nous ne pouvons ignorer les fractures territoriales et numériques, qui privent encore trop de Français d’un accès équitable à la santé. Les déserts médicaux ne sont pas seulement des zones sans médecins : ce sont aussi des territoires où la prévention et l’information sont absentes et où l’accès aux soins devient un parcours du combattant. Je propose donc de créer de tiers lieux de prévention dans ces zones, véritables espaces d’accompagnement, d’information et de soins de proximité. En combinant innovation sociale et mobilisation locale, nous pourrons reconnecter ces territoires au cœur de notre système de santé. Je tiens par ailleurs à attirer l’attention sur un problème essentiel qui menace l’excellence de notre système de santé la diminution alarmante du nombre de spécialistes, notamment en pédiatrie et en psychiatrie. Ces secteurs, si essentiels pour nos enfants et pour les plus vulnérables, ne peuvent être laissés en souffrance. L’excellence médicale française, bâtie sur des décennies de formation rigoureuse et d’expertise reconnue, risque de s’éroder si nous n’agissons pas. Il serait illusoire de croire que nous pourrons maintenir le même niveau de soin et d’accompagnement avec un nombre décroissant de médecins. Certes, la délégation de tâches représente une avancée bienvenue, mais cela ne pourra jamais remplacer la présence, indispensable, de spécialistes compétents, capables de répondre aux besoins complexes de nos concitoyens. Investir dans la formation et l’attractivité de ces métiers, c’est investir dans la santé et l’avenir de notre nation. Mes chers collègues, si les défis sont immenses, notre capacité à les relever l’est aussi. Nous tenons entre nos mains la possibilité d’assurer la pérennité et l’excellence de notre système de santé. Prévention, innovation, accès pour tous : ces priorités doivent guider nos choix. Il est indispensable aujourd’hui d’envisager des réformes structurelles. C’est ensemble que nous trouverons des solutions pour protéger notre modèle social, pour le rendre plus juste, plus durable et plus efficace. C’est ensemble que nous garantirons à chaque Français, où qu’il vive, une santé digne de nos valeurs et de nos ambitions. L’examen de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale constitue une occasion précieuse de poser les bases d’un système de santé plus juste, plus efficient et tourné l’avenir. La parole est à Mme Corinne

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, je concentrerai mon propos sur la branche autonomie de ce PLFSS, dont l’objectif de dépenses pour 2025 s’élève à 42,4 milliards d’euros.

des besoins d’investissement dans les Ehpad, estimé à plus de 7 milliards d’euros à horizon 2030, auxquels il faut ajouter le domiciliaire. Ce sont donc plus de 10 milliards d’euros qui devront, au total, être programmés. Le texte soumis par le Gouvernement, dont nous discutons aujourd’hui, n’apporte aucunement les marges de manœuvre nécessaires

par les professionnels des secteurs de la santé, du social et du médico social. Voilà six ans que les gouvernements successifs nous présentent des écrans de fumée, entraînant une frustration et une colère

définitive, tout cela n’aura été qu’une énième promesse non tenue, qui bafoue de surcroît une proposition de loi adoptée par la représentation nationale. Il y a pourtant urgence à préparer la société à la massification du vieillissement.

réinstaurer un équilibre entre Ehpad publics, Ehpad privés à but non lucratif et Ehpad privés à but lucratif, notamment en taxant les superprofits de ces derniers, comme le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain proposait de le faire le mois dernier, lors de l’examen du texte de notre collègue Jean Luc Fichet. Nous faisons face à un défi majeur, que notre société doit relever. Les enjeux du vieillissement, de la perte d’autonomie, de l’isolement aussi, requièrent des moyens d’ampleur. Avec ce PLFSS, nous passons une fois de plus à côté des vrais sujets dont les Français, y compris les élus, dans tous nos territoires, aimeraient pourtant, très logiquement, que nous

vous l’appelez « contribution de solidarité par le travail ». Ayez au moins le courage de dire clairement que vous demandez aux salariés de travailler une journée gratuitement Alors que certains nous promettaient de travailler plus pour gagner plus, les mêmes nous proposent à présent de travailler plus pour gagner moins… Bien évidemment, nous répondons non ! Il serait profondément injuste de demander de nouveau aux Français de travailler sans être payés. Cela s’appelle du bénévolat. Et je ne connais aucun bénévole dans les entreprises ou dans la fonction publique, car tout travail mérite salaire ! La parole

Si j’approuve l’intention du Gouvernement de réduire les dépenses publiques, je ne peux m’empêcher de penser que l’instabilité fiscale chronique dans les outre mer est un frein au développement. Augmenter le coût du travail, c’est frapper en plein cœur la timide amélioration des chiffres de l’emploi que connaissent certains de ces territoires. Recentrer davantage les exonérations, c’est aussi aller à rebours de ce qu’exigent ces économies.

Or la progression des salaires peut constituer une réponse au problème du coût de la vie, lui aussi structurellement plus élevé. Abaisser les seuils d’exonération reviendrait en réalité à faire des économies en trompe l’œil. L’augmentation des cotisations se traduirait immanquablement par des suppressions d’emplois, ce qui accroîtrait mécaniquement les dépenses sociales – assumées en grande partie par les départements – tout en entretenant le cercle vicieux du chômage. Et je ne parle même pas des emplois qui risquent de basculer dans le secteur secteur informel… Je crois profondément qu’il est temps de chercher des réponses à même de tourner les outre mer vers le développement et de cesser de prendre des décisions par à coups. Cela m’amène à quelques observations sur la méthode. Je suis bien consciente que le Gouvernement a préparé ce projet de loi dans un délai contraint. Mais cela n’apaise en rien mon exaspération de le voir réutiliser la même méthode, que nous décrions régulièrement.

avec l’adaptation par ordonnances, le Gouvernement choisit une fois de plus de priver le Parlement de l’examen des dispositions applicables aux outre mer, en contrepartie d’une concertation. Pour ma part, je considère que les deux sont compatibles : nous pouvons et engager une concertation et débattre au Parlement. L’habilitation demandée à l’article 6 prévoit un délai de six mois, ce qui laisse très peu de temps à la concertation. Je crois, au contraire, qu’il faut se laisser le temps de la discussion pour améliorer durablement ces dispositifs et les stabiliser. Enfin, l’effet rétroactif de l’ordonnance est paralysant pour les employeurs. À l’heure où la délégation sénatoriale aux outre mer, que j’ai l’honneur de présider, conduit une étude sur la coopération régionale, il va sans dire que le coût du travail, face à la concurrence des pays avoisinants,

que l’on ne cède pas au Sénat, serait, elle aussi, affaiblie par la hausse des cotisations. L’augmentation se répercuterait en effet sur les prix, déjà vertigineusement élevés. Malgré son succès touristique, Saint Barthélemy affronte l’émergence de la concurrence venue des autres îles de la Caraïbe, qui se développent sur le même segment touristique. C’est pour cette raison qu’elle bénéficie d’un dispositif d’exonération différencié, qui a notamment contribué à y maintenir le plein emploi, le taux de chômage étant en dessous de 4 %. Je souhaite que ce dispositif soit préservé.

je salue tout d’abord le travail colossal des rapporteurs et leur souci de construire, en responsabilité, le budget de la sécurité sociale, dont le déficit inédit de 18 milliards d’euros nous impose cette année, sans alternative, une trajectoire nette de redressement des comptes sur plusieurs exercices si nous voulons espérer un retour à l’équilibre. L’urgence est donc à l’écriture d’un projet à même de stopper la vertigineuse flèche descendante du déficit depuis 2020 et la période covid. Comme ce PLFSS n’a pas été adopté à l’Assemblée nationale, cette tâche importante incombe au Sénat. Résorber le déficit n’est pas qu’une opération technique. Chaque mesure adoptée aura des conséquences directes sur la vie des Français. Notre commission s’est donné pour cap, sur un chemin étroit et difficile, de répartir l’effort, de protéger l’emploi et les retraites modestes, de soutenir nos hôpitaux ainsi que l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap. Tenir ce cap est essentiel non seulement pour maintenir l’essence même de notre modèle français de protection sociale, envié de par le monde, mais aussi pour répondre à l’évolution des besoins de notre société, aujourd’hui

Je pense, par exemple, au grand âge, aux nombreux efforts qu’il nous reste à faire pour que la prévention et le dépistage deviennent naturels, pour éviter la survenance de maladies et la multiplication de parcours de soins longs et coûteux. Il nous faut certainement, et immédiatement, dépenser moins ; surtout, il nous faut dépenser mieux. Réduire les dépenses, c’est d’abord chercher la justice sociale : que la rectitude budgétaire s’impose à tous, que chacun participe à l’effort collectif. Réduire les dépenses, c’est aussi chercher les poches d’économies et remettre à plat rapidement certains dispositifs qui n’ont pas été révisés depuis longtemps. Réduire les dépenses, c’est encore lutter contre la fraude, repenser et prioriser le contenu du panier de soins, réduire le gaspillage de produits, de pansements, de médicaments non utilisés,

Élue de terrain et de la ruralité, je n’ai de cesse d’être guidée par le souci de l’humain et par l’intérêt général, avec pragmatisme. Je considère l’innovation utilisée à bon escient comme une source d’amélioration de la santé et de gain de temps, d’énergie et d’argent. Généraliser l’intelligence l’intelligence artificielle pour les tâches administratives permettrait aux professionnels de santé, qui y passent près de 30 % de leur temps, de se consacrer davantage à leurs patients. Je plaide également pour davantage de fluidité des parcours de soins et pour la refonte, attendue et annoncée, du statut de l’infirmier, indispensable maillon du système de santé, surtout dans les territoires carencés en médecins.

Enfin, tendre vers un PLFSS équilibré et contenu est aussi l’occasion d’identifier des freins administratifs qui ne sont pas toujours justifiés. L’administration doit participer à l’effort de rigueur, ne serait ce qu’en ne produisant pas de règles compliquées et superflues, et en ayant un rôle de facilitateur du travail des soignants, au service des patients et de l’intérêt général. Face aux crises, les Français n’ont jamais manqué ni de courage ni d’esprit solidaire. Nous devons faire de même !

Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale porte une ambition claire : organiser le redressement de nos comptes tout en préservant notre modèle social. Cette ambition, nous ne pouvons que la partager. À l’occasion de cette discussion générale, permettez moi de rappeler quelques généralités. Selon les données de l’OCDE, la France se classe en tête des pays qui taxent le plus, puisque les prélèvements obligatoires

de ce PLFSS, il vous appartiendra d’engager des réformes structurelles pour retrouver une trajectoire soutenable. La prise en charge de l’autonomie, la réorganisation de notre système de santé et le développement des services de la petite enfance ne peuvent plus attendre. Ces chantiers sont immenses, mais aussi cruciaux. En attendant, si notre commission a partagé l’ambition affichée dans ce texte, nous avons proposé une répartition plus équitable des efforts nécessaires. Il s’agit là d’un choix politique assumé.

a ainsi pris soin de protéger les emplois, en particulier ceux qui correspondent aux salaires modestes, ou encore les petites retraites, tout en répondant aux besoins des hôpitaux, des établissements médico sociaux et des départements.

soutiendra l’aide à domicile et garantira la gratuité des fauteuils roulants, que le Président de la République avait annoncée sans la financer : grâce au Sénat, c’est chose faite. Enfin, la commission a adopté des mesures pour mieux responsabiliser patients et soignants et lutter contre la fraude. Elles portent notamment sur l’incitation des soignants à consulter et alimenter davantage le dossier médical partagé, afin de réduire le nombre d’actes redondants.